La séance est ouverte. Le compte rendu intégral de la séance du mercredi 7 octobre 2020 a été publié sur le site internet du Sénat.

c'est avec tristesse et émotion que nous avons appris la disparition, le 11 septembre dernier, de Christian Poncelet, qui fut sénateur des Vosges de 1977 à 2014 et président du Sénat pendant une décennie, de 1998 à 2008.

lors de cette émouvante cérémonie d'adieu à laquelle assistaient de très nombreux habitants de Remiremont et des Vosges, ainsi bien sûr que de nombreuses personnalités politiques. J'ai salué la mémoire d'un homme de devoir qui portait le gaullisme au plus profond de son engagement. Un homme dont le parcours continuera de marquer le Sénat, le département des Vosges et la commune de Remiremont. Quel destin que celui de Christian Poncelet ! Un destin républicain, car la République ouvre tous les champs du possible à ceux qui, par la puissance de leur travail et la force de leur caractère, se mettent au service de leurs concitoyens. Son père, qu'il perdit très tôt, était mécanicien agricole, et sa mère dut élever seule cinq garçons, auxquels elle transmit le goût du travail et de l'effort. Son grand-père, ancien combattant de la Grande Guerre, lui inculqua le patriotisme, cet amour de la France qui ne le quitta plus. Sa vie fut synonyme de volonté et de courage. Christian Poncelet s'inscrivit à des cours du soir pour acquérir sa qualification de contrôleur aux Postes, télégraphes et téléphones. Il devint agent de la fonction publique et fut promu technicien dans un central téléphonique à Paris. de convictions chrétiennes, Christian Poncelet ressentit très tôt l'envie de mettre son esprit, ses forces et son coeur au service des autres. Il s'engagea au sein de la Confédération française des travailleurs chrétiens, la CFTC, et ce combat lui ouvrit les portes de la politique. Sa rencontre avec Pierre Mendès France joua un rôle déterminant dans son initiation en politique. Ce fut en effet, ainsi qu'il l'a expliqué plus tard, la personnalité qui le marqua le plus après le général de Gaulle. Dès 1958, Christian Poncelet milita au sein de l'Union démocratique du travail, l'UDT, aux côtés de René Capitant, d'Yves Guéna, de Léo Hamon. Leur ambition était alors d'associer justice et efficacité, ordre républicain et mouvement social. Christian Poncelet s'engagea en faveur de l'élection du Président de la République au suffrage universel. Il se présenta à la députation en 1962, il laboura le terrain sans relâche, il sillonna sa circonscription des Vosges, sans cesse à l'écoute des maires. de 34 ans, il devint alors l'un des 233 élus de l'UNR à l'Assemblée nationale. Ce fut le début d'une longue carrière politique au cours de laquelle il ne perdit jamais une seule élection. Les élections cantonales de 1963, puis municipales de 1965, confirmèrent son ancrage territorial dans ce département qu'il aimait tant. Un ancrage qu'il devait à son épouse Yvette, originaire de Saulxures-sur-Moselotte. À partir de 1972, Christian Poncelet enchaîna les secrétariats d'État. Au sein du gouvernement de Pierre Messmer, il fut secrétaire d'État aux affaires sociales, puis au travail et à l'emploi. Il défendit alors la dimension sociale de l'entreprise, il souhaita faire reculer les accidents du travail, il relança aussi l'idée de la participation. Il devint ensuite secrétaire d'État chargé de la fonction publique. Après le décès du président Pompidou, il fut appelé au budget auprès de Jean-Pierre Fourcade dans le gouvernement de Jacques Chirac. Il fut le dernier ministre chargé du budget à avoir présenté un budget en équilibre ! En 1976, il devint président du conseil général des Vosges et appela tous les élus à s'associer à lui, sans esprit partisan. Ce département, il ne cessa de l'incarner. Il fut l'un de ses plus brillants et déterminés ambassadeurs. La diversification de l'économie vosgienne à la suite de la crise de l'industrie textile, l'équipement général du département et de ses communes, ainsi que le désenclavement des Vosges, avec l'arrivée du TGV jusqu'à Remiremont et Saint-Dié et la modernisation du réseau routier transvosgien, portent la marque profonde de son action. 1977, il devint secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement. Mais sa résolution était prise : il souhaitait devenir sénateur des Vosges. Très largement élu, il intégra la commission des finances. Le gaulliste qu'il était siégea au sein du groupe du Rassemblement pour la République, aux côtés de Maurice Schumann et de Charles Pasqua. Au cours de ses premières années de mandat sénatorial, il s'illustra comme rapporteur d'une commission d'enquête sur les difficultés de l'industrie textile, puis d'une mission d'information sur la politique de décentralisation. Il paracheva son ancrage territorial dans les Vosges en étant élu maire de Remiremont en 1983. Trois ans plus tard, il devint président de la commission des finances du Sénat. Il prôna une réduction des déficits, refusa l'augmentation des prélèvements obligatoires et proposa un contre-budget au Gouvernement. Il fut sans cesse à l'écoute de ses collègues de la majorité comme de l'opposition. Au printemps 1998, Christian Poncelet commença sa campagne en vue de la présidence du Sénat. Il se voulut rassembleur et déclina ainsi son slogan : « une présidence modeste au service d'un Sénat ambitieux ». Il fut élu. Le Sénat s'enorgueillit alors d'avoir à sa tête un homme aux origines modestes, ancré dans cette terre des Vosges. Dans l'exercice de ses fonctions de président du Sénat, Christian Poncelet ne cessa de défendre le bicamérisme comme condition de la démocratie. Dès son arrivée, il appela les sénateurs à partir ensemble à la reconquête de l'opinion. Une reconquête qui passait, selon lui, par une attitude responsable lors du vote des lois : « Il ou du toujours oui. » Il plaça la décentralisation, « facteur de libération des initiatives et des énergies locales », au coeur au coeur des débats. Il déclarait : « Il faut donner aux collectivités locales les instruments d'une véritable autonomie, leur conférer de nouvelles compétences, leur reconnaître un pouvoir réglementaire et consacrer leur autonomie fiscale. parfaitement d'actualité ! Sous l'impulsion de Christian Poncelet, la révision constitutionnelle de 2003 permit que les projets de loi « ayant pour principal objet l'organisation des collectivités territoriales » soient soumis en premier lieu au Sénat.

un Sénat capable de développer ses propres capacités d'expertise, de resserrer ses liens avec les collectivités locales et de s'adapter au projet européen. s'attacha à accentuer le suivi sénatorial de la construction européenne en créant notre antenne à Bruxelles et l'association des Sénats d'Europe. Il avait une prédilection pour la diplomatie parlementaire, qu'il tenait pour « un canal de représentation des peuples au plan international ». Il promut le bicamérisme, notamment grâce à l'organisation d'un Forum des Sénats du monde. Longtemps président du groupe interparlementaire d'amitié France-Vietnam- pays dont il se disait « passionné depuis toujours » -, il fut un défenseur inlassable

La présidence de Christian Poncelet fut aussi marquée par des efforts, couronnés de succès, pour mieux faire connaître notre institution. Au-delà d'actions de communication fortes, comme le lancement de la chaîne parlementaire Public Sénat, cette politique d'ouverture s'orienta tout particulièrement vers le monde des entreprises et la mise en place de stages d'immersion en entreprises destinés aux sénateurs. Elle se traduisit également par une politique culturelle, à travers le renouveau du Musée du Luxembourg ou l'organisation

Le 7 mars 2005, il réunit les États généraux de la démocratie locale et de la parité, un sujet sur lequel il s'était engagé. 2003, Christian Poncelet fut élu à l'Académie des sciences morales et politiques. Les symboles qu'il choisit pour orner son épée d'académicien résument

comme son enracinement dans son département d'origine, la mirabelle de Lorraine et la croix de Lorraine, fidélité gaulliste oblige. Pour l'évoquer, ses amis parlent d'un homme de consensus, d'un homme de dossiers, d'un homme de coeur, travailleur et exigeant. Nous garderons de Christian Poncelet le souvenir d'un grand président du Sénat, d'un grand serviteur de l'État, d'un grand parlementaire, d'un élu de proximité profondément attaché à son département des Vosges et à sa commune de Remiremont, et aussi d'un humaniste, d'une personnalité d'une grande simplicité, agréable dans ses relations avec autrui. En ce moment de recueillement et de mémoire, je souhaite renouveler à ses filles, à ses petits-enfants, à ses arrière-petits-enfants, ainsi qu'à toutes celles et tous ceux qui l'ont accompagné tout au long de sa vie, les condoléances sincères de l'ensemble des sénatrices et des sénateurs de la République. J'ai naturellement une pensée pour son J'ai naturellement une pensée pour son épouse, qui nous a quittés il y a plus d'un an. Christian Poncelet restera présent dans nos mémoires

Il a éperdument aimé une terre qui n'était pas celle de sa naissance, et à laquelle il est désormais lié à tout jamais. Comme si, en s'éteignant, sa vie entière nous disait que son destin avait tout fait pour le conduire là ou son coeur a choisi de rester, sans doute parce qu'il portait en lui les desseins d'un idéal plus haut, un idéal secrètement embrassé à sa naissance et auquel il était demeuré intimement lié jusqu'à sa disparition. Enfant, Christian Poncelet fut arraché à ses Ardennes natales et à sa mère par la guerre. Valmy, aujourd'hui El Kerma, et l'Algérie française l'accueillirent. Sa famille alsacienne, qui avait fait le choix de la France en 1870 et qui y résidait, l'y recueillit pendant l'Occupation. Une fois la France libérée par le général de Gaulle, dans les pas duquel il inscrira par la suite son engagement politique, Christian Poncelet effectue son service militaire et aspire à devenir officier de la Légion étrangère : le sens profond de l'autre, le sacrifice, même suprême, inspiraient déjà ses choix, l'intuition, confuse encore mais naissante, que les valeurs de la République seront l'étendard de sa vie entière. Servir toujours, et, dans sa vie, il ne se détourna de cette vocation que brièvement, par amour pour la fille unique d'un menuisier et d'une tisserande, Yvette Miclot, qui deviendra son épouse et à laquelle il ne voulait pas n'offrir qu'une vie d'absences. Il intègre alors l'École nationale supérieure des postes, télégraphes et téléphones, et, même s'il ne s'agissait sans doute pas de son choix de coeur, il était fier de dire, le regard facétieux, qu'il était le produit de l'École des télécommunications, et non celui de l'École nationale d'administration. Sa carrière d'ingénieur, qu'il qualifiait de « raisonnable », l'était sans doute trop pour que se taise l'aspiration au progrès humain et social qui sommeillait en lui. Elle ne suffit bientôt plus à étancher sa soif de « faire » et sa volonté d'oeuvrer à l'amélioration des conditions de travail de celles et ceux avec lesquels il partageait son quotidien. emprunte donc le chemin du syndicalisme et, mû dans son action par ses origines modestes, lui qui était issu d'une famille paysanne porte une attention bienveillante, de chaque instant, aux plus fragiles. En 1953, il fait ses premières armes en animant une grève dure contre le Gouvernement, pour s'opposer à son projet de modification du régime de retraites. Homme du peuple, il le restera lorsque, dix ans plus tard, élu député, il se dit prêt à démissionner quand le général de Gaulle menace de réquisitionner l'armée pour mettre un terme à la grève des mineurs. De cette expérience syndicale, il disait enfin qu'elle n'était certainement pas étrangère à l'une des priorités qu'il avait souhaité mettre en oeuvre en parvenant à des responsabilités gouvernementales : la création de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail. Car le prolongement de l'engagement syndical de Christian Poncelet par un engagement politique devient vite une évidence, et nul chemin ne semble assez escarpé pour le détourner de ce qui devait être sa voie : servir son pays. Il commence à y songer en 1953, profondément inspiré par sa rencontre avec Pierre Mendès France, qui détermine son entrée en politique. Celui qui deviendra son ami l'entraîne un jour dans l'Eure, en pleine campagne électorale, au cours de laquelle il ferraille contre les bouilleurs de cru. Il y perdra son siège, ce dont Christian Poncelet saura en toute occasion se souvenir, lui qui, tout en sachant se montrer ferme et parfois impitoyable, pouvait également manier avec virtuosité le tutoiement et savait convaincre les esprits comme les coeurs. Cette rencontre avec Pierre Mendès France fut également fondatrice de sa volonté farouche d'oeuvrer constamment au dépassement des clivages partisans, avec pour seule considération l'intérêt supérieur de la Nation. Il se disait d'ailleurs libre des considérations politiciennes, comme en témoigne son vote pour François Mitterrand en 1981, 1981, qu'il assumait pleinement. C'est dès 1962 que ce jeune homme de 34 ans se lance dans ce qui sera l'une des plus grandes et des plus longues aventures politiques de la V République, dans le « pays de sa femme », comme il aimait à le dire. Les Vosgiennes et les Vosgiens se prirent immédiatement d'affection pour cet homme chaleureux et simple, un jour de novembre, lorsqu'ils le choisirent pour porter leur voix à l'Assemblée nationale. Le lien qu'ils nouèrent alors devint indéfectible. Jamais il ne sera rompu : dix ans député,

« Je vis les Vosges », disait Christian Poncelet, qui en sillonnait toutes les routes. Entre Charmes et Bussang, Lamarche et Senones, il prenait plaisir à aller dans tous les villages, à la rencontre de cette population qu'il aimait tant, au coeur de ces paysages auxquels il se sentait charnellement lié et qu'il évoquait souvent en parlant aussi de sa passion pour la chasse. Convivial, sans façons, disponible, proche des siens et authentique, si bien qu'il fut bientôt affectueusement surnommé « Ponpon », il était aussi et surtout un homme d'action et de dossiers, qui a profondément transformé sa terre d'élection. Sa mémoire infaillible, sa fine connaissance du territoire et sa fougue étaient saluées de toutes et tous. Il était à la fois un homme de dialogue et d'autorité, de colères tempétueuses et d'écoute pleine d'égards et d'affection. Il était d'ailleurs aussi affable en apparence qu'il savait se montrer dur dans le combat politique. Il exécrait la trahison, dont il avait une conception aussi large que l'importance qu'il accordait à la fidélité et à l'amitié. Son appétit politique se nourrissait de combats face aux adversaires qu'il s'était désignés : Lionel Stoléru d'abord, puis Christian Pierret et enfin Philippe Séguin. De ce caractère singulier, de cette énergie immense, il fit profiter les Vosges en oeuvrant au désenclavement du territoire, à travers le « Y » vosgien, l'aménagement des routes départementales partant vers Saint-Dié, Remiremont et La Plaine, ainsi que l'arrêt du train à grande vitesse à Épinal, Remiremont et à Saint-Dié. Il fut également l'un des artisans majeurs de la conversion économique d'un territoire dépendant de l'industrie textile, auquel il donna une vitalité nouvelle avec l'implantation de nombreuses entreprises portée et soutenue par le conseil général. Les Vosges, mais aussi la France, mais aussi la France, car Christian Poncelet aura également servi avec dévouement et efficacité les gouvernements de Pierre Messmer, de Jacques Chirac et de Raymond Barre. Loyal et compétent, il occupa de hautes fonctions, telles que le secrétariat d'État chargé des affaires sociales, ceux de l'emploi et de la population, de la fonction publique, du budget ou encore des relations avec le Parlement. Le parcours de cet enfant des Ardennes, qui n'avait pas obtenu le brevet, fut forgé par son immense force de caractère ; une page blanche écrite par un autodidacte ambitieux, généreux et travailleur, à l'encre de la méritocratie, ce qui expliquait sans doute pourquoi Christian Poncelet était si peu sensible aux honneurs et aux faveurs. S'il n'aimait pas exhiber titres et succès, il a pourtant à son actif de nombreuses réalisations. Il en évoquait une avec une fierté

Il concevait les responsabilités nationales non pas comme la marque d'une promotion personnelle, mais comme une manière différente de servir son territoire. À aucun instant il n'abandonna la politique locale, lui qui considérait qu'un engagement politique sans enracinement n'avait aucun sens, et qu'il aurait alors ressemblé « à un à un satellite qui avait perdu le contact de la Terre ». Ce contact avec sa terre des Vosges, Christian Poncelet le consolide et le solidifie, en 1977, avec son élection au Sénat. Il aimait d'ailleurs souligner combien l'élection sénatoriale était singulière, parce qu'elle ne dépendait pas uniquement des étiquettes politiques, mais aussi d'une équation personnelle, d'un lien de confiance et d'estime réciproque entre élu et grands électeurs, d'un attachement profond à un territoire. En 1986, il devient président de la commission des finances, ce qui le conduit à la présidence du Sénat, qu'il emporte le 2 octobre 1998, 1998, un siècle après un autre Vosgien, Jules Ferry. Cette présidence ne lui fut pas offerte. Il dut aller la conquérir avec méthode et ténacité, à force d'attentions pour chacune et chacun, dont le souvenir dans cette chambre est impérissable. Parce qu'il fut sincèrement meurtri par les mots d'un ancien Premier ministre, qui parla d'une « anomalie constitutionnelle » en évoquant la Haute Assemblée, il décida de placer sa présidence sous le signe de la défense d'une idée noble du bicamérisme, qui était pour lui la pierre angulaire de la démocratie. Il voulait que le Sénat exerce la plénitude des prérogatives que lui reconnaît la Constitution : il souhaitait qu'il se fasse, au quotidien, la voix des territoires de France et organisa, dans cette perspective, les États généraux des territoires. voyait la décentralisation comme la « seule voie qui conduise à l'esprit d'entreprise », comme l'écrivait le général de Gaulle, qu'il citait alors pour défendre une République territoriale, fruit d'une réforme de l'État et de la gouvernance locale pour que les décisions soient prises au plus près des Françaises et des Français. Il voulait aussi que le Sénat s'ouvre davantage au monde social et économique et aux forces vives de la Nation. Il défendait sans relâche une conception exigeante du rôle du législateur, en prônant un contrôle et une évaluation des politiques publiques toujours plus poussés. Il aspirait également à mieux faire connaître le Sénat des Françaises et des Français, avec les expositions de photographie, que Paris peut encore apprécier au jardin du Luxembourg, et en participant au lancement, voilà vingt ans, de la chaîne Public Sénat. Visionnaire sur ce que devait être l'avenir de la décision publique en France, il ouvrit enfin grand les portes du Sénat aux citoyennes et aux citoyens, à travers l'organisation de rendez-vous citoyens, pour que cette maison de la démocratie soit pleinement la leur. Européen enfin, Christian Poncelet l'était profondément. Lui savait sans doute mieux que quiconque le coût de la guerre, pour avoir dédié sa vie à un territoire lacéré par les conflits. Député européen, il fut un ardent défenseur de la coopération entre les peuples, et un ami de la Chine, précieux pour les relations privilégiées que la France entretenait avec elle. Il se définissait d'ailleurs comme un « Européen convaincu », car il savait sans doute mieux que quiconque que la paix, oeuvre de cette singulière communauté de destin qu'est l'Europe, n'a pas de prix et qu'elle est au coeur même de ce qui est avant tout une manière de penser le monde. Christian Poncelet aura vécu cinquante-deux ans de vie politique, durant laquelle il n'aura jamais connu la défaite. Sa dernière élection au conseil général des Vosges, emportée en 2011 au bénéfice de l'âge, sera son ultime pied de nez à celles ou ceux qui, tout au long de sa vie publique, ont caressé l'espoir de le battre. Sa terre d'adoption le pleure aujourd'hui comme le plus enraciné de ses enfants. « Aimer et avoir la foi », disait-il avec simplicité en parlant du sens de l'engagement de toute une vie au service de Remiremont, des Vosges et de la France. La voix de Christian Poncelet, en cet instant et devant sa famille et ses proches, se confond avec la nôtre et avec celle de la République tout entière. Elle résonnera pour toujours dans cet hémicycle : « Aimer et avoir la foi ». À sa famille, à ses filles, à ses anciens collègues et amis du Sénat, à ses anciens collaborateurs et aux Vosgiens, j'exprime au nom du Gouvernement nos condoléances les plus sincères et le témoignage de notre profonde sympathie. Monsieur le ministre, je vous propose d'observer un moment de recueillement.

La séance est reprise. Mes chers collègues, pour le respect des règles sanitaires, je vous rappelle que le port du masque est obligatoire dans l'ensemble du palais. Il vous est demandé de laisser un siège vide entre deux sièges occupés. L'hémicycle fait l'objet d'un nettoyage et d'une désinfection chaque semaine ; les micros sont régulièrement désinfectés. J'invite chacune et chacun à veiller au respect des distances de sécurité. Je rappelle également que les sorties de la salle des séances devront exclusivement s'effectuer par les portes situées au pourtour de l'hémicycle. Afin de limiter la circulation de documents, vous êtes invités à utiliser vos tablettes et la fonctionnalité « En séance » sur le site internet du Sénat pour prendre connaissance du dérouleur et des amendements. Les conclusions adoptées par la conférence des présidents réunie mercredi 7 octobre sont consultables sur le site du Sénat. En l'absence d'observations, je les considère comme adoptées.- L'ordre du jour appelle la nomination des membres de la commission spéciale chargée du contrôle des comptes et de l'évaluation interne. Conformément aux articles 8 et 103 du règlement, la liste des candidats remise par les bureaux des groupes et le délégué des sénateurs Cette liste sera ratifiée s'il n'y a pas d'opposition dans le délai d'une heure suivant cette publication. Le délégué des sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe a transmis les noms de sénateurs pour siéger au sein de deux commissions permanentes. Conformément à l'article 8 du règlement, ces candidatures ont été publiées. Elles seront ratifiées si la présidence n'a pas reçu d'opposition dans le délai d'une heure.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

Madame la présidente, madame la présidente de la commission des affaires sociales, madame la rapporteure, mesdames, messieurs les sénateurs, la proposition de loi que nous examinons aujourd'hui témoigne de la volonté du Gouvernement d'agir en faveur de l'emploi pour tous. Pour que la relance de notre économie soit la plus inclusive possible, les solutions d'accès à l'emploi doivent être déployées au coeur des territoires. Après l'unanimité obtenue à l'Assemblée nationale, c'est désormais à votre assemblée, celle des territoires, de se prononcer. Je salue l'enrichissement du texte par la commission des affaires sociales du Sénat, et tout particulièrement le travail de Mme la rapporteure Frédérique Puissat. J'en profite pour féliciter Mme Catherine Deroche pour sa récente élection comme présidente de la commission des affaires sociales. La commission a su proposer des outils complémentaires de pilotage des expérimentations, tout en gardant comme boussole l'insertion de nos concitoyens les plus éloignés de l'emploi. La discussion d'aujourd'hui est symbolique à plus d'un titre. Premièrement, elle revêt une grande importance à l'heure où les plus vulnérables peuvent être fragilisés par la crise économique. Cette loi découle directement de la Stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté, annoncée en septembre 2018 par le Président de la République. Elle porte la transcription du Pacte d'ambition pour l'insertion par l'activité économique de 2019, dont elle reprend certaines propositions. Elle prolonge une expérimentation, « territoires zéro chômeur de longue durée », mobilisant les territoires pour proposer des emplois à ceux qui en sont le plus éloignés. Elle s'inscrit dans la philosophie de « France Relance » : tous les leviers doivent être utilisés pour donner un emploi à chacun, aux jeunes, aux seniors, aux moins qualifiés. Elle fait suite à l'annonce d'un dispositif de soutien exceptionnel de 300 millions d'euros en faveur des structures d'insertion par l'activité économique et des entreprises adaptées. Ces orientations budgétaires sans précédent traduisent l'ambition du Président de la République de parvenir à intégrer 100 000 salariés supplémentaires dans les parcours d'insertion et 40 000 autres dans les entreprises adaptées. Deuxièmement, le texte que nous nous apprêtons à étudier a fait l'objet d'une large coconstruction. Dès son élaboration, il a été proposé par des parlementaires et concerté avec les acteurs des structures de l'insertion par l'activité économique et avec l'association Territoires zéro chômeur de longue durée. Pendant sa discussion à l'Assemblée nationale, un travail constructif a été mené par les députés de tous les groupes, majorité comme opposition, qui a permis d'obtenir l'unanimité. Nous pouvons en être fiers. Les débats que nous avons eus ont permis de mieux répondre aux problématiques des personnes les plus éloignées de l'emploi, en oeuvrant à leur insertion et à leur retour durable vers l'emploi. Vous le savez, ce texte renforce deux très beaux outils qui permettent d'appliquer des méthodes complémentaires pour insérer les personnes les plus éloignées de l'emploi. Le titre I est consacré au renforcement du secteur de l'insertion par l'activité économique Le titre II est consacré à la prolongation et à l'extension de l'expérimentation « territoires zéro chômeur de longue durée ». Le titre III est quant à lui un titre de coordination et de mise à jour. jour. L'insertion par l'activité économique est un outil puissant de retour à l'emploi, que cette proposition de loi vise à renforcer. Cette solution d'accès à l'emploi permet d'accompagner le retour à l'emploi de personnes qui en sont durablement éloignées, à partir d'une activité salariée, complétée de formations, au sein d'une structure d'insertion conventionnée par l'État. Pour accompagner et accélérer la consolidation de ce secteur, cette proposition de loi apporte de la simplification pour les structures d'insertion elles-mêmes et de la sécurité pour les personnes en parcours d'insertion. Tout d'abord, elle prévoit un changement nécessaire : la suppression de l'agrément préalable délivré par Pôle emploi et son remplacement par le Pass IAE. la nouvelle plateforme de l'inclusion, les structures d'insertion par l'activité économique pourront recruter sans avis préalable. Elles partageront l'information relative aux personnes qu'elles recrutent directement, sans passer obligatoirement par un tiers prescripteur. Les prescripteurs pourront proposer aussi directement des candidats au recrutement par le biais de la plateforme de l'inclusion. Ce texte permettra donc une simplification des règles de recrutement pour l'ensemble des structures d'insertion par l'activité économique, leur permettant d'embaucher plus rapidement et d'être plus visibles. Cette mesure est attendue de tous et c'est donc une très bonne nouvelle. Dans le même temps, il nous semble nécessaire de prendre en compte la diversité des situations au sein des structures d'insertion par l'activité économique. C'est la raison pour laquelle nous saluons le travail d'écoute de Mme la rapporteure, qui a su entendre les préoccupations des acteurs en vue d'aménager le contrat passerelle et d'y ajouter la possibilité d'un cumul de contrats. Le Gouvernement soutient ces avancées issues du travail de la commission. Dans cette optique, le Gouvernement vous proposera de prolonger une expérimentation en cours dans les entreprises d'insertion par le travail indépendant (EITI), celles-ci constituant la dernière famille des structures de l'IAE. Ensuite, cette proposition Ensuite, cette proposition de loi créait initialement le CDI « inclusion des seniors », qui apporte des éléments de sécurisation pour ces personnes jusqu'à leur retraite. Le Gouvernement proposera de rétablir l'articulation introduite, lors de la discussion à l'Assemblée nationale, entre le CDI « inclusion des seniors » et le contrat à durée déterminée d'insertion (CDDI), notre objectif étant de lutter contre la précarité des seniors. C'est une innovation majeure pour le secteur de l'insertion par l'activité économique, qui, jusque-là, ne proposait que des contrats courts renouvelables jusqu'à concurrence de vingt-quatre mois au maximum. Tout salarié d'une structure d'insertion par l'activité économique (SIAE) de plus de 57 ans au moment du renouvellement de son parcours pourra se voir proposer un CDI, si sa situation ne lui permet pas de retrouver un emploi dans le secteur de droit commun. Ce dispositif remplacera ainsi, pour les plus de 57 ans, les CDDI, qu'il est possible de renouveler par dérogation à partir de 50 ans. Sans trahir la philosophie de l'insertion par l'activité économique, celle du « sas », nous poursuivrons ainsi l'objectif de lutter contre la précarité des seniors éloignés de l'emploi, en en leur permettant d'accéder à un CDI. Dans son titre II, cette proposition de loi vise également à prolonger et à étendre l'expérimentation « territoires zéro chômeur de longue durée

Elle vise à insérer les personnes dans l'emploi en partant de leurs compétences et des besoins des bassins d'emploi. Elle repose sur des CDI à temps choisi. Cette expérimentation, née de la loi du 29 février 2016, adoptée à l'unanimité de l'Assemblée nationale et du Sénat, et soutenue par le mouvement associatif, a rencontré un intérêt certain dans les territoires. Aujourd'hui, treize entreprises à but d'emploi (EBE) existent dans dix départements et emploient 820 personnes, dont 770 personnes privées durablement d'emploi (PPDE), dans le cadre d'un projet collectif utile et complémentaire de l'offre d'emploi préexistante.

Le dispositif consiste à recruter en CDI à temps choisi tous les demandeurs d'emploi volontaires du territoire au chômage depuis plus d'un an sur des activités nouvelles, utiles au territoire et correspondant aux souhaits et aux capacités des PPDE. Je salue le Je salue le travail et la persévérance de Laurent Grandguillaume, président de l'association Territoires zéro chômeur de longue durée, de Michel de Virville et de Patrick Valentin, vice-présidents, et de Louis Gallois, président du fonds d'expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée. Le Gouvernement soutient cette expérimentation prometteuse et est prêt à augmenter la « taille du laboratoire » pour lui permettre de faire ses preuves. Au cours des discussions à l'Assemblée nationale, le Gouvernement a prouvé qu'il savait entendre les préoccupations du terrain et évoluer. Le nombre de territoires pouvant être habilités s'élèverait à soixante, conformément à ce qui a été voté à l'Assemblée nationale. L'engagement du Gouvernement est clair. Ce nombre pourrait être actualisé pour éviter de laisser de côté des territoires qui seraient prêts. Dans le cadre de la navette, comme je m'y étais engagée, nous souhaitons aboutir à la rédaction offrant le plus de flexibilité possible, pour permettre l'habilitation des projets de territoire. Le recours à un texte réglementaire serait susceptible de nous offrir cette souplesse qui répond à l'attente des différents acteurs. Je poursuivrai le travail avec les rapporteurs des deux chambres d'ici à la réunion de la commission mixte paritaire, pour qu'avec les acteurs concernés nous puissions aboutir à une solution respectueuse des territoires et de la volonté des parlementaires. Je le répète, aucun territoire prêt ne doit être laissé de côté. Nous voulons également construire un dispositif responsable au regard des finances publiques. Dans ce cadre, nous saluons l'enrichissement permis par le travail de la commission quant aux dispositifs de suivi de l'expérimentation. À ce stade, la solution issue des travaux de la commission des affaires sociales concernant le financement de l'expérimentation par les départements nous apparaît problématique. Elle fragilise selon nous la position de chef de file des conseils départementaux au titre de leur compétence en matière Cela ne nous semble pas souhaitable. Nous vous proposerons donc de revenir à la rédaction initiale, qui permettait de respecter la compétence du département, mais aussi son expertise et sa connaissance du terrain, en lui laissant le choix de valider ou pas le lancement d'une expérimentation. Faire confiance aux départements, qui sont les acteurs historiques de l'insertion, nous paraît primordial. Je le redis très clairement : aucun projet d'expérimentation ne se fera contre la volonté des départements. Mais la mobilisation d'un département doit logiquement se traduire par sa contribution au financement de l'expérimentation.

l'articulation entre les allégements généraux de charges applicables, depuis 2019, aux cotisations sociales et le mécanisme en discussion. C'est une question d'équité pour les entreprises visées, le III de l'article 7 excluant de son application les structures d'insertion par l'activité économique, ce qui leur permet de jouer leur rôle de sas sans être pénalisées. Sur le terrain, les deux leviers renforcés par les deux premiers titres de cette proposition de loi démontrent déjà au quotidien leur complémentarité. D'un côté, l'insertion par l'activité économique propose un parcours temporaire de retour vers l'emploi et des modalités spécifiques d'accueil et d'accompagnement,

dans les deux cas, une même conviction : le fait de donner un emploi à tous est un facteur essentiel de dignité pour les personnes et de cohésion pour l'ensemble de notre Ces expérimentations sont proches, dans l'esprit, de ce que pourrait être le nouveau service public de l'insertion et de l'emploi, au travers de leur inscription dans un projet de territoire, incarné par les comités locaux pour l'emploi. Mme Brigitte Klinkert, ministre déléguée chargée de l'insertion, sera à mes côtés, dans les semaines qui viennent, pour défendre ce projet de coordination renforcée entre tous les acteurs. Mesdames, messieurs les sénateurs, il s'agit d'un beau texte, utile et nécessaire. Dans cette période d'incertitude et de difficultés accrues pour les plus précaires, son adoption est dans l'intérêt de tous et de tous les territoires. Je n'en doute pas, nous saurons aboutir, dans le respect de nos convictions, à un texte de loi satisfaisant. Vous le savez, la procédure accélérée a été engagée sur ce texte ; nous avons tous à coeur de voir son examen aboutir au plus vite. La commission mixte paritaire aura la responsabilité de travailler à son équilibre définitif.

rapport de Mme Frédérique Puissat, rapporteur de la commission des affaires sociales.

la proposition de loi que nous examinons aujourd'hui porte fortement la marque du Gouvernement, qui a décidé son inscription à l'ordre du jour et a engagé la procédure accélérée. Notons-le, le recours à cette procédure, qui écourte le débat, n'est pas une garantie de célérité. nous avons adopté en urgence, l'été dernier, le dispositif de don de chèques-vacances pour le personnel soignant, qui doit arriver à échéance le 31 octobre prochain, mais dont le décret d'application n'est toujours pas paru Si l'on peut espérer que le présent texte aura davantage de suites, je regrette tout de même que la procédure suivie nous prive d'une étude d'impact ou encore d'un avis du Conseil d'État. Le titre I de la proposition de loi vise à mettre en oeuvre certaines des propositions du pacte d'ambition pour l'insertion par l'activité économique. Ces mesures répondent aux difficultés signalées par les acteurs de terrain ; elles me semblent, pour

Le « Pass IAE », qui s'appuie sur le développement d'une plateforme numérique de l'inclusion- en cours de déploiement -, devrait permettre de fluidifier les recrutements et de supprimer des démarches redondantes. Ce passage à une logique partenariale fondée sur la confiance suppose un contrôle de l'éligibilité des bénéficiaires. Le texte étant muet sur ce point, la commission des affaires sociales a prévu, de manière à répondre aux interrogations des acteurs de terrain, qu'un décret déterminerait les modalités de ce contrôle ainsi que la possibilité, en cas de non-respect de la démarche, de retirer la capacité d'autoprescription à une SIAE. Notre commission a en a en revanche renvoyé à un arrêté, plutôt qu'à un décret, la liste des prescripteurs habilités. La création, à l'article 2, d'un contrat à durée indéterminée (CDI) dit « inclusion senior » répond aux besoins d'un public particulier, pour lequel la logique de tremplin qui sous-tend l'IAE est inadaptée.

la possibilité de déroger, à titre exceptionnel, pour les salariés seniors rencontrant des difficultés particulières, à la durée maximale de vingt-quatre mois de renouvellement des CDD, au-delà de l'âge de 57 ans, en complément du CDI inclusion senior.

ce qui concerne les entreprises de travail temporaire d'insertion (ETTI), la commission a clarifié l'articulation du CDI inclusion senior avec les dispositions législatives relatives au CDI intérimaire. La commission a également apporté des ajustements rédactionnels à d'autres mesures relativement consensuelles introduites à l'Assemblée nationale. En revanche, l'expérimentation d'un « contrat passerelle », permettant à une entreprise d'insertion ou à un atelier ou chantier d'insertion de mettre à disposition, pendant une durée déterminée, sous forme de prêt de main-d'oeuvre à but non lucratif, un salarié en fin de parcours d'insertion auprès d'une entreprise de droit commun, n'est pas accueillie favorablement par certains acteurs de

Pour répondre aux inquiétudes des acteurs de terrain, la commission a précisé le cadre de cette expérimentation, en introduisant, pour les bénéficiaires, une condition d'ancienneté de quatre mois dans un parcours d'IAE, en limitant la durée de la mise à disposition à trois mois renouvelables et en dispensant de période d'essai le salarié en cas d'embauche par l'entreprise utilisatrice. En complément à ce « contrat passerelle », la commission a introduit un dispositif de « temps cumulé », qui vise à permettre une transition progressive entre un contrat d'insertion et un CDI ou un CDD à temps partiel en levant, sous conditions, le seuil de la durée hebdomadaire de travail au sein des SIAE, De la même manière, il sera possible de déroger, dans le cadre de ce dispositif, au minimum de vingt-quatre heures hebdomadaires en contrat à temps partiel de droit commun. Dans son deuxième volet, cette proposition de loi vise à prolonger de cinq ans et à étendre de dix à soixante territoires l'expérimentation « territoires zéro chômeur de longue durée ». Cette expérimentation consiste à permettre l'embauche de chômeurs de longue durée en contrats à durée indéterminée, pour des tâches non couvertes par l'économie de marché. Les emplois ainsi créés sont presque intégralement financés par les pouvoirs publics, en faisant l'hypothèse que le retour à l'emploi permet à la collectivité d'éviter des dépenses directes et indirectes à hauteur du coût assumé pour les financer. Cette Cette expérimentation suscite de nombreuses attentes. J'ai pu mesurer à quel point l'association porte ce dispositif et je me permets de saluer l'engagement de tous les bénévoles et de tous les élus locaux, qui ont à coeur de défendre leur vision. J'ai pu échanger de manière constructive avec eux tout au long de mes travaux.

apporter une vraie réponse à la problématique de l'exclusion nécessite sans doute d'augmenter les moyens que nous consacrons à cette politique. En effet, celle-ci peut être vue comme un investissement social et l'absence de neutralité financière ne doit pas être un obstacle à la poursuite de l'expérimentation. La question que nous devons nous poser est donc celle de l'efficience du dispositif « territoires zéro chômeur de longue durée » par rapport à celle d'autres outils de la politique de lutte contre l'exclusion, notamment les structures d'insertion par l'activité économique. À cet égard, l'expérimentation menée depuis 2016 permet de tirer de premiers enseignements, dont il convient de tenir compte pour la suite. À ce jour, elle a permis d'embaucher un peu moins de 1 000 personnes, sur les 4 000 personnes privées d'emploi potentiellement éligibles. Cette montée en charge plus lente que prévu s'explique en partie par les difficultés rencontrées par les porteurs de projet, qui soulignent la nécessité d'accompagner chaque projet territorial et, sans doute, de trouver des financements complémentaires, au moins pour la période de démarrage des entreprises à but d'emploi. Je considère donc qu'il s'agit d'un début encourageant. Les évaluations réalisées montrent que la situation matérielle et morale des personnes embauchées s'est nettement améliorée, ce qui confirme, s'il en était besoin, qu'il est préférable d'occuper un emploi stable que d'être en situation d'exclusion. Le comité scientifique, qui doit rendre son rapport final dans les semaines à venir, semble conclure que l'on n'observe pas encore d'effets positifs notables pour les territoires eux-mêmes, mais il est sans doute trop tôt pour tirer des conclusions à ce sujet. À la différence des structures d'insertion par l'activité économique, les entreprises à but d'emploi proposent des contrats à durée indéterminée et ne se donnent pas pour objectif explicite l'insertion dans l'emploi de droit commun. Ce facteur semble décisif pour permettre la stabilisation dans l'emploi des personnes embauchées, en supprimant l'épée de Damoclès que représente la fin prévue du contrat. Pour autant, l'expérimentation comporte, de ce fait, ce que le comité scientifique appelle un « impensé », qui touche à l'évolution professionnelle des personnes embauchées. Sans doute faudra-t-il remettre en question ce parti pris, qui n'est d'ailleurs pas partagé par tous les porteurs de projet, et mettre davantage l'accent sur la formation de ces personnes, dans une logique de parcours vers l'emploi. L'expérimentation montre également que la concertation entre les acteurs locaux permet de développer des activités nouvelles, utiles aux territoires. Si le critère de non-concurrence avec le secteur marchand semble globalement respecté, une attention particulière devra être portée à l'articulation avec les acteurs de l'insertion par l'activité économique. Il faudra aussi se demander si, à moyen terme, l'absence de perspective d'évolution professionnelle et salariale dans les EBE n'est pas de nature à créer des frustrations et s'il n'existe pas un risque d'effet d'éviction par rapport à certains emplois du secteur marchand qui présenteraient un niveau supérieur de contraintes tout en étant rémunérés au même niveau. Enfin, l'un des éléments les plus intéressants, à mes yeux, de cette expérimentation réside dans la logique de territoire sur laquelle repose le dispositif. Plutôt que d'appliquer des règles administratives parfois inadaptées aux réalités de terrain, on fait confiance, au travers de ce dispositif, à la capacité des acteurs locaux de dépasser les cloisonnements et de travailler ensemble pour chercher des solutions.

Au-delà de la question du coût, de nombreux points d'amélioration existent et certains éléments amènent à s'interroger sur les présupposés de la démarche. La poursuite de l'expérimentation permettra d'approfondir ces réflexions. Elle doit donc concerner un nombre limité de territoires

qui ne doit pas se limiter à apprécier l'opportunité d'une pérennisation ; il s'agira par exemple de se demander si le modèle des entreprises à but d'emploi peut trouver sa place parmi les autres outils de la politique de l'emploi et s'il convient de le cibler sur certains publics ou sur certains territoires aux caractéristiques spécifiques. Les évolutions législatives proposées par rapport à la loi de 2016 sont marginales. Les améliorations attendues devront donc être mises en oeuvre dans les textes réglementaires d'application, d'une part, et dans la gouvernance du dispositif, d'autre part. La proposition de loi prévoyait initialement de rendre obligatoire la participation des départements au financement de l'expérimentation. Aujourd'hui, tous les départements comprenant un territoire expérimentateur participent au financement des emplois créés, à un niveau variable mais généralement faible. le principe d'une participation obligatoire pose plusieurs difficultés, du fait notamment que l'on ne connaît pas son montant, les modalités de calcul étant renvoyées à un décret sur lequel nous n'avons, à ce stade, aucune information. Tant que le dispositif demeure expérimental, il représente une ligne marginale du budget de la politique de l'emploi et de l'insertion, et l'on et l'on pourrait être tenté de donner satisfaction à toutes les prétentions de ses promoteurs. Les louanges que l'on pourrait ainsi récolter ne me semblent pour autant pas justifier le fait que nous nous abstenions de jouer notre rôle de législateur. La commission des affaires sociales a donc choisi de s'inscrire pleinement dans la démarche expérimentale, en précisant, entre autres choses, les objectifs de l'expérimentation et de son évaluation. Pour finir, je dirai quelques mots du titre III, qui contient diverses mesures liées de près ou de loin à l'emploi et à l'insertion. Une disposition censurée de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020, concernant l'articulation du bonus-malus sur les contrats courts avec les allégements généraux de cotisations sociales, a refait son apparition. La commission l'a supprimée, afin de réaffirmer son opposition au bonus-malus et pour tenir compte de la concertation en cours sur la réforme de l'assurance chômage. Conformément à la position habituelle du Sénat, elle a également supprimé les demandes de rapport. En revanche, elle a adopté les articles 8 et 9 , qui prévoient la prolongation de deux autres expérimentations, afin de pouvoir disposer du recul nécessaire pour en apprécier la pertinence, ainsi que l'article 9 , qui crée une expérimentation du contrat de professionnalisation en portage salarial. La parole

Avec la crise sanitaire, ces chiffres sont amenés à s'aggraver. Le creusement des inégalités est de plus en plus préoccupant. Près de 15 % des Français restent sous le seuil de pauvreté. Ces dernières années sont marquées par une stagnation des revenus les plus faibles, avec l'un des plus longs arrêts de la progression du niveau de vie jamais enregistrés depuis la Seconde Guerre mondiale. Pour contrer ce phénomène, les politiques de redistribution et d'insertion représentent l'un des plus puissants leviers contre la pauvreté. Être sans emploi ne constitue pas un destin, ce n'est pas une fatalité. Toutes les initiatives sont précieuses en matière de politique d'insertion. C'est pourquoi le groupe Les Indépendants soutient pleinement la proposition de loi que la Haute Assemblée examine à présent. Au-delà de ce soutien, nous avons aussi déposé des amendements visant à l'améliorer, à apporter une pierre supplémentaire à l'édifice, afin que chacun puisse retrouver le chemin du travail dans les meilleures conditions possible. Le titre I porte sur le dispositif d'insertion par l'activité économique. En 2020, l'État a investi 1 milliard d'euros dans l'insertion par l'activité économique, qui associe mise en situation professionnelle, accompagnement personnel et formation.

Nous sommes d'accord avec ce principe et c'est bien l'objet de cette proposition de loi. Il nous semble néanmoins qu'il est important que Pôle emploi garde un certain contrôle sur les renouvellements de contrats, au-delà des vingt-quatre premiers mois ; il s'agit, rappelons-le, de situations exceptionnelles. L'accès à la formation doit également être amélioré et ne pas être de l'ordre du virtuel. Enfin, pour les mêmes raisons, nous devons renforcer l'évaluation et le suivi des bénéficiaires dans le temps, pour permettre notamment la comparaison de ce dispositif avec les autres actions qui s'adressent à un public similaire. Le travail de la commission des affaires sociales a permis d'évoluer en ce sens. Le titre II porte sur le dispositif expérimental « territoires zéro chômeur de longue durée », lancé par ATD Quart Monde. L'idée est intéressante ; au lieu de subventionner l'inactivité,

Le principal débat porte sur le ciblage et le coût du dispositif. Effectivement, l'inspection générale des finances et l'inspection générale des affaires sociales préconisent de recentrer le dispositif davantage sur les bénéficiaires du revenu Rappelons-le, il s'agit de contrats à durée indéterminée, contrairement aux dispositifs d'insertion par l'activité économique, qui sont des dispositifs de transition. Il paraît opportun de réserver ces créations d'emploi aux personnes les plus éloignées de l'emploi, ce qui ne semble pas être le cas actuellement.

de vue du coût, les entreprises à but d'emploi restent déficitaires. Nous ne pouvons pas encore nous prononcer sur la viabilité financière de l'expérimentation à long terme ; c'est pourquoi des évaluations plus solides sont nécessaires. Je souhaite à présent vous présenter un amendement tendant à proposer un dispositif d'insertion complémentaire, dont le département de l'Allier est l'initiateur. Il s'agit de permettre aux bénéficiaires du RSA de reprendre une activité partielle dans une entreprise, à hauteur de 15 heures par semaines, tout en continuant à percevoir leur allocation pendant un an. À l'issue de cette durée, les salariés concernés pourraient bénéficier d'un contrat initiative emploi, subventionné par le département. Il s'agit d'une sortie en douceur, incitative mais sécurisée, du dispositif du RSA. Nous savons que plusieurs départements seraient intéressés par une telle expérimentation. C'est pourquoi, en complément de cet amendement, nous avons également déposé aujourd'hui une proposition de loi visant à lancer cette nouvelle expérimentation, qui n'appartient à aucun parti, si ce n'est à celui du bon sens et du progrès social. Chers collègues, je vous invite à vous associer à cette démarche. Nous pensons que, au Sénat, il est important de permettre aux collectivités territoriales d'innover, d'expérimenter de nouvelles solutions dans leurs domaines de compétence. Le groupe Les Indépendants - République et et le rapport de Mme Frédérique Puissat, rapporteur de la commission des affaires sociales. Ce texte contribuera à enrichir les actions des pouvoirs publics en direction des personnes en situation de vulnérabilité économique, bien souvent associée à une vulnérabilité sociale.

Le dispositif « territoires zéro chômeur de longue durée » est novateur, ambitieux et dynamique. Il répond tant aux besoins des demandeurs d'emploi de longue durée qu'aux besoins non satisfaits de nos territoires,

amener à nous interroger sur la perception, très française, des fameux « indicateurs de performance ». À Pierre Cahuc, qui évoque « le coût des emplois créés », à partir d'un calcul qui mériterait un débat, nous opposons non seulement le coût de la privation d'emploi, dont l'ampleur a été confirmée par une étude réalisée par le département d'économie de l'Université libre de Bruxelles, mais également l'utilité écologique et sociale de cette expérimentation. nombre des activités supplémentaires créées dans les dix territoires expérimentateurs ont trait à la transition écologique et permettent la sauvegarde de l'environnement. Il convient dès lors d'en tenir compte et de mesurer, par exemple, leur impact sur notre empreinte carbone.

Ce sont ces activités, qui visent à l'amélioration de « nos patrimoines critiques, à savoir notre patrimoine naturel et la santé sociale », pour reprendre la formule de la sociologue Dominique Méda, que nos fameux indicateurs économiques de performance devraient impérativement prendre en compte, en s'appuyant sur les nouveaux indicateurs de richesse introduits par la loi du 13 avril 2015 issue

nous n'avons pas le temps d'attendre ! Or, plutôt que d'aller dans ce sens, la commission des affaires sociales du Sénat a décidé de modifier sensiblement le dispositif, mettant à mal l'opérationnalité de ses dispositions. C'est, selon mon groupe, regrettable. Le Sénat va donc mettre à mal ce consensus, se faisant, au passage, le porte-voix des détracteurs, minoritaires, de l'expérimentation. Peut-être le jeu en aurait-il valu la chandelle si le Sénat avait souhaité être plus ambitieux, afin de permettre à un plus grand nombre de territoires qui sont prêts et capables de répondre au cahier des charges de se lancer, mais il n'en est rien. Bien au contraire, le texte que nous examinons cet après-midi prévoit d'imposer une double tutelle et un copilotage : premièrement, une tutelle de Pôle emploi sur le choix des personnes qui pourront être recrutées dans les entreprises à but d'emploi ; deuxièmement, une tutelle des directions sur le choix des activités développées par ces entreprises ; enfin un copilotage des préfets avec les comités locaux. Ces tutelles vont vider le projet de ses fondamentaux, en faisant reposer celui-ci sur un principe de défiance et en recentralisant la démarche. cette défiance est l'antithèse du droit à l'expérimentation, mais elle va également à l'encontre d'un principe dont le Sénat se fait régulièrement le défenseur : faire confiance à l'intelligence territoriale, faire confiance aux territoires. Territoires présentera donc des amendements de suppression de ces mesures, afin de revenir au texte de l'Assemblée nationale. C'est seulement s'ils sont adoptés que nous pourrons voter ce texte. La parole

Le droit à l'emploi constitue donc un droit fondamental, et il incombe au législateur d'en garantir l'effectivité pour nos concitoyens. Malgré les différentes réformes structurelles mises en place par les gouvernements successifs, 4,2 millions de personnes sont aujourd'hui éloignées de l'emploi, dont 2,7 millions depuis plus d'un an. Nous partageons donc le constat des auteurs de la proposition de loi : nous n'avons pas tout essayé pour lutter contre le chômage. Il appartient au législateur de s'appuyer notamment sur le tissu associatif pour parvenir à des évolutions concrètes en vue de ramener vers l'emploi les personnes qui en sont privées. La crise sanitaire inédite que nous traversons constitue un choc économique et social de grande ampleur. Un certain nombre de secteurs l'ont subi de plein fouet ; je pense notamment au commerce, à l'hôtellerie et à la construction. En avril dernier, en plein confinement, nous assistions à une hausse inexorable du taux de chômage, atteignant son plus haut niveau depuis vingt-cinq ans. Le nombre de demandeurs d'emploi a ainsi augmenté de 22,6 %, ce qui représente plus de 840 000 personnes. Nous le savons, les jeunes sont les premiers touchés par les effets de la crise. Ils sont plus de 700 000 à être arrivés sur le marché du travail et le contexte sanitaire laisse à penser que bon nombre d'entre eux éprouveront des difficultés en matière d'insertion je pense en particulier aux jeunes les moins qualifiés, qui seront le plus exposés au chômage et à la précarité. Devant cette réalité, le Gouvernement a déjà annoncé un certain nombre de mesures, dans le cadre du plan France Relance. débloqués 300 millions d'euros en faveur des structures d'insertion par l'activité économique et des entreprises adaptées, avec un objectif de 100 000 salariés supplémentaires dans les parcours d'insertion. Pour compléter ces dispositifs, l'État doit être aux côtés des acteurs économiques, des collectivités territoriales et des associations. L'insertion par l'activité économique constitue ainsi une riposte efficace, qui concilie l'économique, le social et le territorial. Le dispositif « territoires zéro chômeur de longue durée », promu à l'origine par des acteurs associatifs de terrain et lancé officiellement en 2016, grâce à une proposition de loi de Laurent Grandguillaume, est une réussite ; les premiers chiffres nous le démontrent.

proposé de l'étendre et d'en faire bénéficier de nouveaux territoires frappés par le chômage. L'expérimentation sera ainsi prolongée de cinq ans et cinquante territoires de plus seront concernés. Cette expérimentation, novatrice en ce qu'elle part des territoires et des compétences des personnes privées d'emploi, offre une solution complémentaire des politiques de l'emploi qui existent dans notre pays. En tout état de cause, nous saluons la vision et les objectifs de cette proposition de loi. Celle-ci met en oeuvre un certain nombre de propositions du pacte d'ambition pour l'insertion par l'activité économique, remis voilà un an au Gouvernement et qui a pour objet de mobiliser, aux côtés de l'État, l'ensemble des acteurs de l'inclusion, les collectivités et les entreprises, dans un esprit de coconstruction. Supprimer la procédure obligatoire d'agrément de Pôle emploi préalablement à toute embauche dans le cadre d'un parcours d'insertion apparaît nécessaire pour faciliter l'entrée dans un tel parcours. C'est pourquoi nous saluons cette disposition. Nous défendrons, à cet égard, un amendement visant à prévoir le passage par un prescripteur habilité, afin de prolonger les parcours dans l'insertion par l'activité économique des salariés en insertion, en lieu et place de Pôle emploi uniquement.

L'expérimentation du contrat de travail renforcé à durée indéterminée, instauré à l'article 3 de la proposition de loi, valorisera une démarche partenariale entre les collectivités territoriales, les entreprises et Pôle emploi, réunis dans un même objectif : l'insertion durable dans l'emploi des bénéficiaires de ce dispositif. Le groupe RDPI soutiendra un certain nombre d'amendements à ce texte. Nous souhaitons en effet permettre à toutes les SIAE, et pas seulement à celles de moins de 50 salariés, de développer la formation, indispensable à la montée en compétences des personnes en parcours d'insertion. Nous défendrons également un amendement visant à mettre en oeuvre la mesure de revalorisation de la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle prévue dans le cadre du plan France Relance. Je conclurai en reprenant les mots inspirants du président du Conseil de l'inclusion dans l'emploi : « L'inclusion n'est ainsi pas l'affaire des exclus : elle est l'affaire de tous, pour redonner à ceux qui sont devenus des " invisibles " une place à part entière dans la société. » Il est donc essentiel de favoriser le partenariat et d'associer l'ensemble des acteurs : entreprises, associations, collectivités territoriales. Tel est l'objet de la proposition de loi, et c'est la raison pour laquelle nous la soutiendrons.

comme la priorité absolue des dix-huit prochains mois. Nous ne pouvons que nous en féliciter dans le contexte actuel. L'ampleur de la crise sanitaire a, en effet, fortement affecté le marché de l'emploi. Après une baisse en trompe-l'oeil pendant le confinement- un grand nombre de personnes sans emploi ayant interrompu leurs recherches -, le taux de chômage devrait grimper à 9,7 % en fin d'année. Avec la reprise de l'épidémie, l'Insee n'exclut pas qu'il atteigne 10 %, alors même que notre pays connaît, depuis près de cinquante ans, un chômage de masse, que les différentes politiques de l'emploi peinent à enrayer. Dans ces conditions, la proposition de loi dont nous débattons aujourd'hui revêt une importance particulière. Je pense, bien sûr, à son premier volet, qui reprend le pacte d'ambition pour l'insertion par l'activité économique et s'inspire de la volonté du Président de la République de faire passer le nombre des bénéficiaires de l'insertion par l'activité économique de 140 000 à à 240 000. La suppression de l'agrément préalable par Pôle emploi ou la mise en place d'un CDI inclusion pour les seniors sont des mesures qui vont dans le bon sens. Je pense surtout à la prolongation de l'expérimentation « territoires zéro chômeur de longue durée ». Je salue ce dispositif, né dans les années 1990 et relancé par ATD Quart Monde il y a près de dix ans pour en finir avec le chômage de longue durée. Il repose en fait sur une idée assez simple : l'embauche en CDI de chômeurs de longue durée payés au SMIC par le développement d'activités locales un fonds financé par la réaffectation des dépenses liées au traitement du chômage. Certains, à l'époque, ont qualifié ce projet de farfelu, voire d'utopique. Mais les grandes réalisations ne sont-elles pas d'abord une utopie ? Le bilan de la première phase est positif : à la fin de l'année 2018, l'expérimentation avait permis à 1 112 personnes de sortir de la privation d'emploi. Malgré tout, plusieurs voix s'élèvent pour reprocher au projet d'être un gouffre financier. la rapporteure elle-même estime que, si le dispositif « propose une réponse novatrice et intéressante à la problématique de l'exclusion », il « représente un coût pour les finances publiques » qui rendrait, à date, « sa généralisation difficilement soutenable ». Mais ce dispositif ne doit pas s'apprécier seulement à l'aune de son aspect financier. Comme l'a rappelé le président du Comité scientifique d'évaluation de l'expérimentation, « l'enjeu prioritaire consiste à ramener à l'emploi les personnes qui en ont été durablement privées et d'apprécier l'impact positif du dispositif sur ces personnes, leur entourage, et plus généralement sur les territoires d'expérimentation La première phase expérimentale a, en effet, montré comment des femmes et des hommes qui allaient très mal ont retrouvé un sens à leur vie et une utilité sociale. Le film de Marie-Monique Robin, qui a

de l'absence d'emploi sur la santé. La perte d'un travail et la difficulté à en retrouver un dégradent la santé des chômeurs : stress, perte de sommeil, problèmes cardiovasculaires, addictions, diabète, dépression ... Selon une étude de l'Inserm, 10 000 à 14 000 décès seraient ainsi imputables au chômage chaque année. C'est pourquoi nous nous réjouissons de l'extension de cette expérimentation, même si les modalités retenues nous paraissent trop restrictives, qu'il s'agisse du nombre de territoires concernés ou de la durée de la prolongation. Certes, les débats à l'Assemblée nationale ont permis de porter à cinquante le nombre de nouveaux territoires, mais cela nous semble encore bien insuffisant. Nous savons que le conseil d'administration de l'association Territoires zéro chômeur de longue durée et déjà validé 122 projets en vue de la deuxième étape. Tous ceux qui remplissent les conditions devraient pouvoir accéder au dispositif. Madame la ministre, vous avez assuré à nos collègues de l'Assemblée nationale qu'il serait possible de rediscuter de ce seuil dans deux ou trois ans. Dont acte Par ailleurs, les territoires qui auront besoin de trois ans pour se préparer disposeront de moins de cinq ans pour expérimenter le dispositif, ce qui est dommageable. Nous regrettons, enfin, certaines orientations prises par notre commission des affaires sociales, s'agissant notamment de la suppression du concours obligatoire des départements au financement des emplois supplémentaires créés, du copilotage du préfet ou de la double tutelle. Ces modifications nous semblent antinomiques de l'esprit de l'initiative, qui repose essentiellement sur la confiance faite aux territoires pour identifier les personnes privées d'emploi et les besoins non satisfaits. Pour ces raisons, nous serons particulièrement attentifs aux débats et au sort réservé aux amendements déposés, notamment ceux du groupe RDSE.

Madame la présidente, mesdames les ministres, mes chers collègues, en 2016, le groupe CRCE avait voté en faveur de l'expérimentation « territoires zéro chômeur de longue durée soutenue par de nombreuses associations, tout en rappelant que seule une politique publique ambitieuse apporterait une solution globale. Depuis 2016, le contexte a été profondément bouleversé par la crise sanitaire due à la pandémie de la covid-19 et, surtout, par ses conséquences économiques, 800 000 personnes supplémentaires au chômage étant venues s'ajouter aux 2 millions de personnes déjà éloignées de l'emploi avant le déclenchement En cinq ans, sur dix territoires, 420 personnes ont pu bénéficier de l'expérimentation et sortir du chômage de longue durée, ce dont nous ne pouvons que nous réjouir, même si c'est un tout petit pas au regard de l'ampleur du phénomène. les initiatives locales ne peuvent remplacer une politique de l'emploi ambitieuse, permettant à chacune et chacun d'évoluer dans sa vie professionnelle, selon ses aspirations, sans perte de revenu et sans jamais passer par la case « chômage ». C'est ce que soutient le groupe CRCE au travers de sa proposition de sécurité d'emploi ou de formation. Dans le cadre d'un nouveau service public de l'emploi et de la formation, auquel toute personne ayant achevé sa scolarité serait affiliée de droit, chacune et chacun pourrait alterner périodes de travail salarié et périodes de formation rémunérées, grâce à une réduction générale du temps de travail rendue possible par les gains de productivité qu'apportent les nouvelles technologies. Ce n'est malheureusement pas la voie empruntée par le Gouvernement, qui, dans son plan de relance de 100 milliards d'euros, n'a prévu que 200 millions d'euros pour le soutien aux personnes précaires. Autrement dit, 0,2 % des crédits du plan de relance sont destinés à assurer la cohésion de la Nation en luttant contre la précarité.

Le Gouvernement prétend sortir les personnes de la précarité, objectif que nous soutenons complètement, mais sa majorité propose, au travers de l'article 7, de supprimer l'application du bonus-malus sur les cotisations d'assurance chômage en cas de recours abusif à l'emploi de courte La droite sénatoriale va encore plus loin, en faisant disparaître tout malus pour les contrats courts. Autrement dit, les employeurs sont invités à recruter en contrat précaire, y compris les seniors, pour lesquels est créé un CDI au rabais. Les personnes auront le choix, désormais, entre la précarité en dehors de l'emploi et la précarité dans l'emploi ... Avec ce texte, c'est la nature même du secteur de l'inclusion par l'activité économique et des expérimentations « territoires zéro chômeur qui est remise en cause. Mes chers collègues, nous savons toutes et tous que la persistance du chômage de longue durée ne relève pas d'abord d'une responsabilité individuelle et qu'elle résulte du système économique et social, ce qui entre forcément en contradiction avec l'article 8, qui prolonge l'expérimentation du renforcement des contrôles sur les chômeurs dans leur recherche d'emploi, et avec l'article 9, qui vise à responsabiliser les salariés l'utilisation de leur compte personnel de formation avant toute prise en charge financière les régions ou Pôle emploi. La droite sénatoriale pense que le cumul des contrats d'insertion et des contrats à temps partiel de moins de 20 heures va permettre de sortir les personnes de la précarité. Ce n'est pas notre avis.

Madame la présidente, mesdames les ministres,

Le 7 octobre dernier, le journal titrait : « Un million de nouveaux pauvres d'ici à fin 2020 ». Ce sont désormais plus de 10 millions de Français qui vivent au-dessous du seuil de pauvreté. La rapporteure du texte à l'Assemblée nationale, Mme Verdier-Jouclas, souhaitait voir dans l'ouverture de la session parlementaire par l'examen de ce texte un « symbole fort adressé à l'ensemble de nos concitoyens touchés par la privation d'emploi ». Je partage son analyse. de la crise que nous traversons, les choix ont un sens. Que nous examinions en ouverture de session la proposition de loi relative au renforcement de l'inclusion dans l'emploi par l'activité économique et à l'expérimentation « territoires zéro chômeur de longue durée la traduction des préoccupations de nombreux Français, la traduction de nos préoccupations. Le symbole est d'autant plus fort que le coeur du texte émane directement du terrain, plus précisément de notre riche tissu associatif.

de construction des solutions localement et elle bat en brèche la logique bien trop souvent descendante de la production de la loi. Les symboles ont toutefois leurs limites. Si les attentes peuvent être grandes à l'égard du texte qu'examine aujourd'hui notre assemblée, soulignons d'emblée que celui-ci n'a pas vocation à supprimer le chômage de masse. Il nous faut prendre en compte les limites et les apports de l'expérimentation. Sur les dix territoires d'expérimentation prévus par la première loi relative aux « territoires zéro chômeur de longue durée » de 2016, 918 personnes ont été embauchées. Étendre le dispositif à cinquante nouveaux territoires ne permettrait que de multiplier approximativement par cinq ce chiffre. C'est donc une goutte d'eau au regard des 2 685 000 chômeurs de longue durée comptabilisés au deuxième trimestre de 2020. Comme Mme la rapporteure Frédérique Puissat l'a indiqué en commission, il s'agit de proposer « une solution complémentaire aux autres outils existants, qui serait particulièrement pertinente pour certains publics ou pour certains territoires L'extension de l'expérimentation ouvre ainsi la possibilité de réaliser un travail sur mesure, au plus près du terrain, tout en posant des jalons nécessaires dans la refondation de la politique de l'emploi. À l'inverse et de manière complémentaire, le plan de relance présenté à la rentrée vise à agir vite et fort pour l'emploi. À titre d'exemple, 1 milliard d'euros sont consacrés à la formation des salariés en activité partielle et au renforcement des compétences. Pour aider les jeunes arrivant sur le marché du travail, le Gouvernement prévoit aussi une enveloppe de 6,7 milliards d'euros, soit un triplement des moyens alloués à l'emploi des jeunes. Enfin, avec la généralisation de l'accompagnement de l'activité partielle, ce sont 9 millions de salariés qui n'auront pas été privés de leur emploi en 2020. Le plan de relance ajoute 7,6 milliards d'euros en faveur de l'activité partielle de longue durée. Avant d'entrer dans le détail du contenu des articles, je souhaite féliciter notre rapporteure, Frédérique Puissat, pour son travail méthodique, mené dans un contexte bien particulier entre la situation sanitaire que nous connaissons et le renouvellement partiel du Sénat, la préparation de ce texte n'a pas été aisée. La majorité de nos collègues n'a pas pu réellement s'imprégner de son contenu, qui ne se limite pas, bien au contraire, à la seule extension de l'expérimentation « territoires zéro chômeur de longue durée ». Les dispositions qui se rapportent à celle-ci sont d'ailleurs reléguées au sein du titre II de la proposition de loi. J'en viens au titre I. Il contient divers dispositifs visant à mettre en oeuvre plusieurs propositions du pacte d'ambition remis au Gouvernement à la rentrée 2019, après concertation avec les acteurs de l'insertion par l'activité économique. Selon la promesse du Président de la République, 100 000 salariés supplémentaires doivent intégrer les parcours d'insertion. L'article 1 est une mesure d'assouplissement, issue de remontées du terrain. Il vise à supprimer l'agrément obligatoire de Pôle emploi pour les embauches au sein des structures de l'insertion par l'activité économique. Il est essentiel de faire confiance aux acteurs locaux. Cet article y contribue.

Certains acteurs de l'IAE ne sont pas favorables à l'expérimentation d'un « contrat passerelle » et demandent avant tout plus de souplesse, plus de confiance en leurs compétences et plus de moyens financiers. Un CDI « inclusion senior » permettrait néanmoins de mieux répondre aux besoins des personnes en fin de carrière. Les amendements présentés par Mme la rapporteure améliorent sensiblement le texte de ces articles.

Grâce à un financement de l'État, ces dernières offrent aux personnes éligibles volontaires un emploi correspondant à leurs compétences, dans le cadre d'activités socialement utiles qui n'entrent pas en concurrence avec le tissu économique local. le texte issu de l'Assemblée nationale a été bonifié. Je salue le passage de quarante à soixante du nombre de territoires ouverts à l'expérimentation, ainsi que la sécurisation des dix premiers territoires et de leur financement. Faut-il accroître davantage le nombre de territoires concernés, alors que 120 territoires seraient déjà candidats ? Je me rangerai à l'avis de Mme la rapporteure entre le coût du dispositif et les externalités positives attendues, la neutralité financière de l'expérimentation n'est pas encore pleinement démontrée. Aussi élargir davantage l'expérimentation tendrait-il à fragiliser l'ensemble du dispositif,

Pour conclure, il est indéniable que le retour en emploi entraîne une amélioration significative de la situation des bénéficiaires, qui retrouvent ainsi une place dans la société et l'estime d'eux-mêmes, tout en voyant un certain nombre de leurs difficultés matérielles se réduire.

« territoires zéro chômeur de longue durée » s'articule parfaitement avec d'autres composantes de l'insertion par l'activité économique. C'est peut-être là une de nos divergences, madame la rapporteure.

Le chômage est une véritable calamité pour notre pays : endémique depuis des décennies, il a été accentué, ces derniers mois, par un confinement forcé qui n'en finit toujours pas pour certaines professions, notamment pour les restaurateurs et cafetiers des Bouches-du-Rhône. Les catastrophiques décisions gouvernementales ne vont faire qu'ajouter la crise économique à la crise sanitaire. Quand des millions de Français auront plongé dans la pauvreté, croyez-vous que notre système de santé en sera renforcé ? Allez regarder ce qui se passe dans les pays pauvres ! Allez voir comment la population y est soignée ! Protéger l'économie et les emplois, mesdames les ministres, c'est protéger nos hôpitaux, donc sauver des vies. Ce sont évidemment les déclassés et les plus fragiles de notre société qui font les frais de la situation actuelle. Un salarié en insertion sur cinq a vu son contrat prendre fin pendant le confinement. Il est donc primordial, en parallèle du plan de relance et des lois de finances pour 2021, de parler d'inclusion et d'honorer le troisième terme de notre devise de notre devise nationale : la fraternité. Le dispositif que vous nous proposez n'a de sens que si l'on applique la priorité nationale. La proposition de loi omet volontairement cette dimension de l'accès à l'emploi pour les Français d'abord. Il ne s'agit pourtant que de solidarité nationale, et donc de justice sociale. Occupons-nous des nôtres d'abord ! Nous n'allons pas prendre à notre charge toute la misère du monde quand 10 millions de Français survivent désormais au-dessous du seuil de pauvreté et 6 millions, dans la réalité, sont au chômage. Je vous le dis, mes chers collègues, pas un seul étranger de plus ne doit être mis à notre charge tant qu'un seul de nos compatriotes sera dans la pauvreté ! Occupons-nous des Français honnêtes et travailleurs, laissés pour compte de la mondialisation sauvage et de la concurrence déloyale ! Ce n'est évidemment pas la direction que prend le Gouvernement, puisque Marlène Schiappa propose d'accorder prioritairement un emploi aux « choufs », c'est-à-dire aux guetteurs des réseaux de trafic de drogue. Après la préférence donnée aux étrangers pour l'emploi la discrimination positive, voilà la priorité aux crapules ... Il s'agit là sans doute de la nouvelle méritocratie républicaine en marche ! On ne peut qu'encourager le recours aux dispositifs favorisant le retour à l'emploi, surtout dans les zones désindustrialisées. Néanmoins, votre dispositif paraît, sous certains aspects, tenir plus du maquillage des chiffres du chômage que d'une politique volontariste de retour à l'emploi. La durée des contrats d'insertion passant de vingt-quatre à soixante mois et celle des contrats à durée déterminée d'usage à plus de cinq ans sont deux points qui m'inquiètent. De nombreux travailleurs vont se trouver précarisés. Or, depuis la crise sanitaire, on voit que les intérimaires, les salariés modestes, tous ces travailleurs qui ont souvent été en première ligne pendant le confinement se retrouvent à la limite de la pauvreté. Il n'y aura plus de chômage de longue durée quand nous aurons recouvré notre souveraineté économique et migratoire pour relocaliser, nous protéger et nous libérer. Vous parlez d'inclusion, mais la mondialisation, c'est la loi du moins cher et du plus fort ; c'est la loi de l'exclusion ! Ces remarques étant faites, je partage évidemment l'impératif de retour à l'emploi des chômeurs de longue durée et voterai

s'explique par un constat partagé : le chômage est une injustice sociale et un fléau national, que la puissance publique doit combattre activement, sans jamais tomber dans le fatalisme, car la priorité des priorités est la politique de l'emploi. Loin des envolées lyriques ou des caricatures méprisantes qui voudraient qu'il suffise de traverser la rue pour trouver du travail, cette expérimentation destinée à la recherche d'emploi est pragmatique. Elle repense l'action publique au service des chômeurs de longue durée. Cette approche est fondamentale. Le rapport sénatorial sur les chiffres du chômage l'a démontré : plus il y a de chômeurs de longue durée, plus il est difficile de faire baisser le chômage durablement ; plus une personne reste éloignée du marché du travail, moins elle a de Entre bénéfice social et équation financière, ce dispositif met en lumière l'échec de la logique de compensation sociale du chômage de longue durée par des aides de toutes sortes, financées par une fiscalité sur le travail toujours plus pesante, sans succès pour l'emploi., l'emploi., le dispositif ne devrait pas coûter très cher, puisque l'État économise autant en prestations sociales et en coûts indirects supportés par la solidarité nationale. surtout à un objectif concret : redonner une chance, une dignité, un élan économique et social à une personne durablement éloignée de l'emploi. Si jamais un désaccord se fait jour au Parlement, c'est évidemment sur le périmètre,

Sachez que, dans mon département, la communauté d'agglomération du pays de Grasse et la métropole Nice-Côte d'Azur sont volontaires. Cette expérimentation serait la bienvenue dans les Alpes-Maritimes, tant pour les élus que pour les entreprises et la population. Par ailleurs, si l'heure est au contrôle et à l'évaluation, nous ne pouvons pas écarter d'un revers de main les critiques de plusieurs rapports, qui soulignent des carences budgétaires et une réalité éloignée de la théorie. C'est la raison pour laquelle je veux rendre hommage au travail pragmatique de Mme le rapporteur, qui, au travers des auditions qu'elle a menées et des déplacements qu'elle a effectués, a cherché à adapter au mieux ce dispositif sur les territoires. Dès lors, je pense qu'une évaluation parlementaire une mission d'information serait opportune, afin de pouvoir rendre le dispositif toujours plus efficient, même si, d'un point de vue budgétaire, après trois lois de finances rectificatives et un plan de relance, le Gouvernement a décidé de faire sauter tous les compteurs, nom du fameux « quoi qu'il en coûte ». Plusieurs réformes antérieures ont été lourdement critiquées pour leur coût. Je pense notamment au CICE. Cependant, l'effondrement économique et social est un péril beaucoup plus grave et imminent, pour les Français, que la dette. Au regard de l'ampleur de la crise, il faudra certainement aller plus loin, plus vite, et encourager la généralisation du dispositif à l'échelle nationale. Le président de la région des Hauts-de-France l'a dit : « nous l'avons expérimenté, et ça marche Pourquoi ne pas aller, demain, vers une régionalisation du dispositif, là où il a été expérimenté avec succès ? Cela signifie que la période de contrôle et d'évaluation devra être resserrée, car, je vous le rappelle, entre l'annonce de l'extension du dispositif, érigée en priorité dans le cadre du plan de lutte contre la pauvreté présenté en septembre 2018 et le vote d'aujourd'hui, il se sera tout de même écoulé plus de deux ans. De nouveaux territoires sont prêts pour l'expérimentation, et les collectivités locales volontaires sont les mieux placées pour raccourcir le chemin vers l'emploi, ajuster les mesures et témoigner des besoins sur le terrain. telle généralisation, qui est une demande fondée, sera la reconnaissance par l'État de l'implication des collectivités locales sur le front de l'emploi. Elle ne devra pas trop tarder, au risque d'éteindre les énergies dans les territoires. Enfin, alors que l'Assemblée nationale a commencé l'examen des crédits du plan de relance, la discussion de ce texte est aussi l'occasion de rappeler que c'est avant tout par le travail que la France remboursera ses dettes et retrouvera le chemin de la croissance. Bien évidemment, le groupe Les Républicains suivra les propositions et la position de Mme le rapporteur.

Madame la présidente, mesdames les ministres, mes chers collègues, la proposition de loi que nous examinons cet après-midi est porteuse d'espoir est porteuse d'espoir et attendue par toutes celles et tous ceux qui oeuvrent à faire de l'inclusion une réalité, afin que toute personne en capacité de se rendre utile à la vie de la cité puisse être accueillie et accompagnée dans ses aspirations.

viable et à visage humain. Permettez-moi d'ancrer mon propos dans la réalité de mon territoire. Depuis 2016, la commune de Pontchâteau, en Loire-Atlantique, est engagée dans la démarche. À l'époque, j'avais assisté à l'une des premières réunions du comité local pour l'emploi. Comme vous le savez, ce comité réunit en même temps les porteurs locaux du projet et les futurs bénéficiaires, dans un dialogue constructif et bienveillant. Tous oeuvrent avec les mêmes préoccupations, en ayant à l'esprit les particularismes territoriaux, en vue de créer une entreprise à but d'emploi et de l'activité. et de l'activité. De ce comité local se dégage une énergie forte et transpartisane, soutenue par l'envie d'essayer ce qui ne l'a pas encore été. Depuis son lancement, le comité local a travaillé, réfléchi, défini son périmètre de mission. Les femmes et les hommes qui le constituent, que j'ai de nouveau rencontrés voilà quelques semaines, ont gardé cette envie. Aujourd'hui, les énergies sont décuplées par la perspective de l'extension de l'expérimentation. Pour autant, j'ai aussi entendu exprimer quelques inquiétudes, inspirées légitimement par le travail parlementaire. En première lecture, l'Assemblée nationale a voté un texte fortement empreint de l'esprit de la loi adoptée sous le quinquennat précédent,

Là où nous voulons tout essayer, quitte à bousculer les approches, vous préférez, mes chers collègues, surcontrôler, encadrer et, finalement, freiner les énergies des chômeurs et des chômeuses. Avez-vous oublié que, à terme, dans ces entreprises à but d'emploi, il y aura des femmes et des hommes aux parcours de vie marqués, hachés, empêchés par un handicap ou des obstacles indépendants de leur volonté ? Samedi 17 octobre 2020, journée mondiale du refus de la misère, alors même que la Banque mondiale prévoit que la pauvreté s'intensifiera

Fine connaisseuse de notre maison, elle saura faire montre de ses qualités de modératrice pour animer et pondérer les débats dans notre hémicycle. Je lui adresse tous mes voeux de réussite et d'épanouissement dans ses nouvelles fonctions Les différentes observations sur la conjoncture économique et la situation actuelle de l'emploi font froid dans le dos. D'après de récentes prévisions de l'Unédic, pas moins de 900 000 emplois sont appelés à être détruits sur l'ensemble de l'année 2020 en France. La pandémie est venue considérablement aggraver le problème du chômage de longue durée, symbolisé par le dépassement, cette année, de la barre des 4 millions de chômeurs relevant de la catégorie A. Selon une étude réalisée en 2015 par l'association ATD Quart Monde, le chômage coûte à l'État 43 milliards d'euros chaque année, dont 15 milliards d'euros de manque à gagner en impôts et en cotisations sociales.

handicap ou à faible qualification. L'Aisne, mon département, souffrait au premier trimestre de 2020 d'un taux de chômage de 11 %, très nettement supérieur à la moyenne nationale. Quatre de ses zones d'emploi figurent parmi les trente le plus durement touchées par le chômage dans notre pays. On y compte 13 000 bénéficiaires du RSA, dont environ la moitié retournent chaque mois à l'emploi. En tant que président de la maison de l'emploi et de la formation de Laon, je suis sensible à cette problématique particulièrement importante. C'est donc avec joie que j'accueillerai l'extension du dispositif « territoires zéro chômeur de longue durée ». En effet, quoi de plus volontariste qu'une politique publique ayant fait ses preuves et visant à opérer un transfert des coûts du chômage, qui relèvent des dépenses passives, vers des dépenses actives d'investissement dans le retour à l'emploi La flexibilité introduite dans le dispositif, s'agissant notamment de la suppression de l'agrément obligatoire par Pôle emploi, est bienvenue pour fluidifier les procédures d'embauche dans les entreprises à but d'emploi et responsabiliser les travailleurs. Une action concertée entre les services publics de l'emploi, les entreprises à but d'emploi du secteur de l'économie sociale et solidaire et le département permettra non seulement aux publics les plus précarisés de remettre le pied à l'étrier, mais aussi, dans une perspective plus large, de recréer une dynamique de cohésion et de renforcer le lien entre citoyens et institutions. Je me dois cependant d'émettre quelques réserves sur certains volets du texte. Par bien des aspects, celui-ci révèle que, en dépit de ses promesses renouvelées de décentralisation, le Gouvernement semble avoir bien du mal à lâcher la bride et à accorder véritablement aux collectivités territoriales la marge de manoeuvre qu'elles demandent. Cela fait trois ans que l'on nous parle d'accélérer la décentralisation, que l'on nous dit que la gouvernance des politiques publiques peut et doit véritablement passer par l'échelon local, afin d'en augmenter l'efficacité et la plus-value pour nos citoyens.

Par ailleurs, il est primordial que nous prêtions aujourd'hui la plus grande attention à ce que le financement du dispositif « territoires zéro chômeur de longue durée » ne se solde pas purement et simplement par l'ajout d'une nouvelle charge publique relevant de la seule responsabilité des départements. Sur la base du rapport établi par la commission, seuls 26 % des salariés embauchés dans les entreprises à but d'emploi percevaient antérieurement une allocation du type du RSA. Ainsi, contraindre les départements à financer l'intégralité des emplois créés grâce au dispositif reviendrait, ni plus ni moins, à tirer sur l'ambulance. Je veux également alerter les défenseurs du projet sur les tensions qui affectent déjà le budget de nombreux départements. Dans l'Aisne, le coût du chômage atteint 114 millions d'euros : plus de 71 % des dépenses de fonctionnement sont dédiées au seul financement des minima sociaux. égard à la diminution des subventions de l'État, solliciter une nouvelle contribution en faveur des politiques de l'emploi semblerait donc peu raisonnable, voire malvenu, et ne ferait que créer une macrocéphalie de ce poste de dépense, au préjudice des autres domaines de l'action publique locale.

L'accent mériterait en outre d'être mis sur le rôle et la participation des intercommunalités, dans la mesure où celles-ci assument déjà la compétence emploi et développement économique. En somme, l'arbitrage que nous devrons

tout particulièrement à ce que la mise en oeuvre du dispositif n'impose pas une concurrence malvenue aux divers organismes déjà déployés dans les territoires et actifs dans la politique de l'emploi. Ainsi, pour ce qui concerne le contrat passerelle, il semble nécessaire de rappeler qu'un certain nombre de dispositifs existants, tels les groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification, ou les périodes de mise en situation en milieu professionnel, ont déjà fait leurs preuves. Les chiffres parlent d'eux-mêmes : en 2018, 70 % des contrats conclus dans le cadre des GEIQ avaient conduit à l'obtention d'un emploi et près de 60 % à l'obtention d'un emploi durable. Il est donc nécessaire que la mise en oeuvre de ce dispositif aille encore plus loin dans la logique de responsabilisation des demandeurs d'emploi. Élever le niveau et la qualité des formations proposées et en diversifier l'offre seront des moyens renforcés pour maintenir les jeunes dans les territoires, raviver l'attractivité et le dynamisme de ceux-ci et former de la main-d'oeuvre spécialisée et qualifiée pour de potentiels futurs bassins d'emploi. À un contexte économique et socioprofessionnel tendu, il est urgent de répondre par des projets d'action sociale ambitieux. Si le projet « territoires zéro chômeur de longue durée » semble sur la bonne voie, il reste encore à lui accorder les moyens financiers et techniques nécessaires pour lui donner toutes les chances de réussir, de pouvoir enfin déployer, à terme, une politique sociale digne de ce nom. À ce titre, je suivrai la position de la commission. La parole

atteint son plus bas niveau depuis dix ans. Depuis le début de la crise, le Gouvernement est mobilisé pour protéger les emplois, les entreprises et les salariés. Tel est le sens des trois projets de loi de finances rectificative, qui ont permis d'engager

territoire candidat à l'expérimentation « territoires zéro chômeur de longue durée » ne reste sur le bord de la route. J'aurais souhaité pouvoir vous présenter l'amendement permettant de

pour permettre aux personnes les plus éloignées de l'emploi de trouver une réponse à leur situation dans le contexte très difficile que nous connaissons. Je ne peux pas laisser dire que nous ne consacrerions que 200 millions d'euros aux personnes les plus fragiles.

simplement de permettre que les entreprises d'insertion par l'activité économique, qui par nature recourent à des contrats

Selon nous, le contrôle, même, doit demeurer un contrôle public, afin d'éviter d'éventuels conflits d'intérêts entre plusieurs structures privées. Mme la ministre du travail a affirmé à nos collègues députés que, demain, grâce à cette précision inscrite dans le texte, le diagnostic pourra être établi soit par des prescripteurs habilités, dont Pôle emploi, soit par les structures d'insertion par l'activité économique

qui sera mis en place dans le cadre de la plateforme de l'inclusion, à des fins de sécurité juridique. Il prévoit notamment le suivi des parcours dans l'insertion par l'activité économique et des aides pouvant être versées dans ce cadre. Il vise également également à étendre la gamme des conséquences éventuelles d'un manquement d'une structure d'insertion par l'activité économique au processus de prescription d'un parcours en IAE, en ajoutant la possibilité de limiter

la possibilité, pour une structure d'insertion par l'activité économique, de recruter directement une personne remplissant les critères d'éligibilité. À l'alinéa 10 de l'article sont évoquées des modalités d'appréciation et de contrôle par l'administration,

un amendement visant à prévoir le passage par un prescripteur habilité, afin de prolonger les parcours dans l'insertion par l'activité économique des salariés en insertion, en lieu et place de Pôle Dans la mesure où la prolongation de ces contrats d'insertion doit rester une exception, le passage par un prescripteur habilité devrait permettre d'offrir au salarié en insertion la possibilité d'étudier, avec l'aide d'un tiers spécialisé, les solutions alternatives ou complémentaires disponibles pour la réussite de son parcours d'insertion. Il s'agit donc d'une mesure de simplification.

Il s'agit de prévoir l'articulation entre les CDI inclusion senior et le renouvellement de contrats à durée déterminée d'insertion (CDDI) en associations intermédiaires (AI) pour les salariés de plus de 57 ans.

à 57 ans du CDDI au CDI senior ; l'employeur garde la main. Il s'agit aussi de maintenir les deux dispositifs

l'avis de la commission ?

Cet article introduit en séance publique à l'Assemblée nationale un amendement du Gouvernement prévoit de mettre en place l'expérimentation d'un « contrat passerelle » permettant la mise à disposition d'un salarié en insertion auprès d'une entreprise de droit commun en vue de son éventuelle embauche. La quasi-totalité des acteurs du secteur de l'insertion est très fermement opposée à ce contrat passerelle. Selon eux, le dispositif proposé ne remplit pas l'objectif de sécurisation des parcours d'insertion permettant de sortir les personnes notamment parce qu'il déstabilise les dispositifs existants pour les associations intermédiaires et pour les entreprises de travail temporaire d'insertion. C'est pourquoi il est proposé de supprimer cet article. Quel est l'avis

l'avis du Gouvernement ? Il y a eu concertation, un pacte a été remis ; cette expérimentation offre un outil juridique souple qui peut devenir un nouveau déclencheur d'embauche, du fait du lien entre SIAE et entreprises ordinaires, et permettra de sécuriser la période de transition professionnelle.

autre qu'une structure d'insertion par l'activité économique. Cette expérimentation doit avoir pour objet exclusif de faciliter le recrutement de personnes en fin de parcours d'insertion par les entreprises de droit commun. Il ne faudrait pas en effet créer, avec ce contrat passerelle, une nouvelle marche avant l'entrée dans un hypothétique emploi durable. Afin de répondre aux mêmes objectifs que ceux du contrat passerelle en évitant ses écueils, nous avions proposé, en commission, de prévoir la possibilité d'un cumul entre un contrat d'insertion et un contrat de droit commun à temps partiel, que la rapporteure a elle-même introduite à l'article 3 A nouveau. Puisque Mme la rapporteure a souhaité conserver, en complément de cette nouvelle mesure, le contrat passerelle, celui-ci doit absolument s'accompagner de garanties pour éviter des effets d'aubaine et une utilisation dévoyée du dispositif. Il s'agit ainsi d'éviter que ce nouveau contrat ne soit assorti d'aucune obligation pour l'entreprise utilisatrice et crée de ce fait un effet d'aubaine. Nous proposons donc, premièrement, que la mise à disposition soit considérée comme une réelle promesse d'embauche et qu'elle soit limitée à quatre que la période de mise à disposition comporte une période d'essai plus longue que celle que prévoit le droit commun, pour permettre à l'utilisateur de vérifier les compétences du travailleur. Vous l'avez compris, mes chers collègues : nous sommes contre la création du contrat passerelle, mais nous avons parfaitement conscience

la commission ?

CDI ou CDD à temps partiel. Ce contrat mixte est censé permettre à la salariée ou au salarié de continuer à bénéficier de l'accompagnement de la structure d'insertion par l'activité économique tout en accomplissant une transition progressive vers l'emploi de droit commun. Faut-il rappeler ici que les structures d'insertion par l'activité économique ont pour objectif d'offrir aux personnes sans emploi un tremplin vers l'économie classique que, par conséquent, il n'est pas nécessaire de cumuler plusieurs contrats ? Nous sommes véritablement en désaccord avec l'idée que la transition du parcours d'insertion par l'activité économique vers le secteur marchand justifierait de déroger au droit commun, en l'espèce au minimum hebdomadaire.

par les contrats à temps partiel sont majoritairement des femmes. En effet, selon une étude de la Direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques de juillet 2020, 31 % des femmes occupent un emploi à temps partiel, et 78 % des 18,4 % de salariés du secteur privé travaillant à temps partiel sont des femmes. Dès lors, ces dérogations auront pour conséquence de renforcer la précarité des salariés, et en particulier des femmes, plutôt que de faciliter la transition vers un contrat de travail classique. Pour toutes ces raisons, nous demandons la suppression de cet article. Quel

à des personnes en parcours d'insertion. C'est une mesure attendue notamment par les conseils départementaux. Elle contribue à rappeler le rôle central des départements en matière d'insertion : ils sont des partenaires essentiels pour l'accès à l'emploi. La PMSMP est une pratique d'accompagnement très demandée, qui a fait ses preuves. Il faut l'élargir et permettre d'y recourir rapidement en élargissant la liste de ses prescripteurs aux conseils départementaux

et de faciliter le parcours du bénéficiaire. C'est un véritable outil pour l'accès à l'emploi

de longue durée » en cours depuis 2017 dans mon département, le Calvados, plus précisément à Colombelles, près de Caen. L'entreprise à but d'emploi, atypique, a été créée en avril 2017.

que de personnes disponibles pour les accomplir. Ce n'est pas l'argent non plus qui manque, puisque, chaque année, le chômage de longue durée entraîne de nombreuses dépenses et manques à gagner. C'est une expérimentation profondément novatrice par son objectif, sa méthode et son financement. Elle améliore la situation des personnes et des territoires, à Colombelles comme ailleurs. C'est pourquoi je suis très favorable non seulement à sa prolongation pour cinq ans, mais aussi à son extension à de nouveaux territoires.

Un département peut ainsi refuser de financer le dispositif et ne pas mettre en place cette expérimentation sur son territoire. Ce dispositif illustre donc plutôt la confiance du législateur et du Gouvernement à l'égard du département et de sa capacité de faire

L'implication du département doit être financière afin d'assurer la protection de ses compétences et de sa capacité à choisir ce qui est le mieux pour son territoire. Les collectivités territoriales veulent être responsabilisées et demandent davantage de compétences pour pouvoir exercer cette responsabilité. Il serait donc dommageable d'empiéter sur les compétences historiques du département en rendant son financement volontaire. Rendre compte de ses choix est essentiel. C'est ce que l'on souhaite pour le département, et cela implique obligatoirement un financement à cet échelon.

en permettant aux acteurs locaux de participer pleinement au pilotage du dispositif au sein des comités locaux pour l'emploi. En effet, les différentes expériences de création de ces comités ont permis d'engager un dialogue constructif avec l'ensemble des acteurs locaux. Ce dialogue vise à préciser les règles de fonctionnement de l'expérimentation en matière de développement des activités et d'embauche, en prenant en compte les spécificités locales. Les entrepreneurs, les chambres consulaires, les centres sociaux, les structures de l'insertion par l'activité économique, les associations, les élus et les habitants doivent rester au coeur du dispositif

voté à l'Assemblée nationale prévoyait un financement obligatoire du fonds d'expérimentation par les départements concernés par le dispositif. Cette obligation de financement a été supprimée sur l'initiative de la rapporteure de la commission des affaires sociales. De notre point de vue, elle doit être rétablie pour ne pas obérer l'extension de l'expérimentation « territoires zéro chômeur de longue durée ». Cet amendement ne tend pas à créer de dépense supplémentaire, puisque ce financement vient se substituer aux prestations déjà

Par ailleurs, l'expérimentation repose depuis son origine sur les initiatives locales. La réussite des projets passera par l'implication de tous les acteurs locaux, sans exception.

territoriale contre le chômage de longue durée est financé « par l'État, les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale, les groupes de collectivités territoriales et les organismes publics

La participation financière sera définie par les textes d'application, en concertation, évidemment, avec les conseils départementaux et l'ADF. Aujourd'hui,

peuvent d'ailleurs être des bénéficiaires du RSA. Dans ce cas, les gains attendus de l'expérimentation doivent être largement supérieurs à la charge induite, le coût lié au RSA étant réduit d'autant. C'est en quelque sorte une stratégie d'économie par l'efficacité de l'action publique, un investissement gagnant-gagnant : gagnant pour le citoyen qui retourne vers l'emploi ; gagnant pour la collectivité qui réduit ses dépenses d'allocation. Pour avoir été présidente de conseil départemental, je sais, comme vous, mesdames,

J'insisterai particulièrement sur la suppression de l'obligation de financement des départements concernés par le dispositif. Cette expérimentation constitue pourtant une vraie réponse face à la crise sociale. Rappelons que l'on attend 300 000 chômeurs supplémentaires d'ici à la fin de l'année. Les collectivités territoriales, particulièrement les départements, acteurs centraux de l'action sociale, doivent soutenir ces projets. La philosophie de l'expérimentation « territoires zéro chômeur de longue durée » implique que les collectivités susceptibles de tirer un bénéfice

à refuser que les départements contribuent de manière obligatoire, dès lors qu'ils sont concernés, me surprend donc. En disant ceci, je vais peut-être

Je suis très favorable à la participation des départements, mais pas par obligation. Je pense qu'il faut les inciter,

En effet, la philosophie du projet implique que les collectivités territoriales susceptibles de tirer indirectement ou directement un bénéfice financier des embauches contribuent effectivement au financement de l'expérimentation.

des suites qu'il convient de donner au projet, la commission des affaires sociales du Sénat me semble avoir considérablement dévoyé l'esprit initial du texte. L'évaluation réalisée par le comité scientifique doit surtout permettre d'analyser les conditions de pérennisation du projet d'expérimentation.

pour bien mesurer les incidences positives, qui doivent peser dans la décision publique, laquelle ne saurait être régie par le seul coût financier à court terme ou une comparaison avec d'autres dispositifs,

Il est indispensable que les élus locaux puissent participer à l'élaboration des travaux du comité scientifique.

Les activités développées dans le cadre de la première phase de l'expérimentation « territoires zéro chômeur de longue durée » présentent des spécificités intrinsèques à la philosophie même de ce projet, mais qui ne se retrouvent plus du tout dans la rédaction que nous propose Mme la rapporteure pour les alinéas

il s'agit bien de répondre à une demande sociale locale qui n'est pas remplie, parce qu'elle n'est pas assez lucrative pour le secteur marchand : tel est le fondement des EBE.

est non pas de contrôler les embauches, mais de permettre à tous les volontaires une sortie de la privation durable d'emploi. Parmi les enseignements tirés de la première étape expérimentale, il est apparu que, pour assurer les fonctions confiées au CLE,

Mais cette expérimentation s'inscrit dans une autre perspective : celle de l'implication des citoyens et des bénéficiaires eux-mêmes aux côtés des collectivités dans la détermination d'une politique adaptée aux spécificités de leurs territoires. expérimentation ont aussi montré combien ce dispositif permettait de recréer de l'entraide et de la solidarité, en favorisant une nouvelle dynamique économique et sociale, sans parler du développement de nouvelles activités liées à la transition écologique, l'aide aux personnes, ou encore la médiation sociale. À ma connaissance, aucun autre dispositif ne propose une forme de démocratie participative plus avancée que celle-là ni ne constitue, parallèlement, un tel approfondissement de la décentralisation. Notre assemblée promeut depuis des années une plus grande confiance dans les collectivités, défend une décentralisation plus importante, mais aussi plus « sur mesure » en fonction des situations locales. Aussi, je suis particulièrement surprise que la commission ait introduit dans le texte un assemblage de dispositions qui traduisent une défiance envers les acteurs locaux et réinstaurent une tutelle des services de l'État sur le dispositif.

mais nous ne pouvons pas accepter que les autres territoires qui se sont investis sérieusement pour répondre au cahier des charges soient empêchés de mener cette expérimentation. C'est pourquoi nous souhaitons qu'elle soit enclenchée dans soixante territoires et que tous ceux qui sont prêts à s'y engager puissent y être intégrés au fur et à mesure. Cela permettra Cela permettra aussi de lever toute interrogation sur les critères de choix d'un territoire ou d'un autre. Mesdames les ministres, nous avons bien entendu votre engagement à ce sujet ; nous resterons donc très attentifs à ce qu'il en soit bien ainsi.

Ce qui pose problème, c'est bien l'ajout du préfet dans le copilotage de l'expérimentation. Alors que nous sommes en train de débattre d'un dispositif qui, par nature, rend possibles d'autres fonctionnements, on observe de vieux réflexes centralisateurs. Il est indispensable que l'expérimentation puisse continuer à être menée au plus près du terrain, en faisant confiance au territoire. C'est pourquoi, au travers de cet amendement,

Notre commission des affaires sociales a souhaité ajouter le préfet dans le copilotage de l'expérimentation. Or il nous semble indispensable que celle-ci puisse continuer à être menée au plus près du terrain, en faisant confiance au territoire. Aussi, au travers de cet amendement, nous proposons de supprimer cette rédaction adoptée par la commission, qui porte un message de défiance à l'égard des territoires.

l'avis du Gouvernement ?

Faute de pouvoir faire figurer dans le texte une garantie que tous les projets territoriaux arrivés à maturité puissent intégrer l'expérimentation, nous souhaitons au moins pouvoir assurer à ceux qui auront été retenus une durée d'expérimentation de cinq ans effectifs. Cet amendement vise donc à prévoir que la durée de cinq ans d'expérimentation sera glissante pour les territoires entrant au fil de l'eau dans le dispositif TZCLD. Ainsi, leur projet pourra se déployer dans de bonnes conditions et sur une durée suffisamment longue pour leur permettre une réelle effectivité et les rendre donc efficaces.

relatif à l'expérimentation territoriale visant à supprimer le chômage de longue durée et, plus précisément, à celles de cet article 5, qui crée un fonds d'expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée. Ce dispositif est le fruit d'une réflexion lancée de façon expérimentale en 2016 ; cette expérimentation a suscité en Corse, région au tissu économique fragile, un écho favorable et un intérêt évident. Plusieurs intercommunalités, des élus locaux, ainsi que le président de l'Assemblée de Corse ont engagé un travail de terrain qui mérite d'être pérennisé l'activation de ce fonds. Ainsi, la Corse pourra disposer de l'appui et de l'accompagnement nécessaires à la lutte contre le chômage de longue durée.

et la mise en oeuvre de la démarche « territoires zéro chômeur longue durée » rencontre des difficultés structurelles. Il est ainsi proposé de garantir que l'expérimentation puisse s'adapter aux spécificités de la collectivité territoriale de la Corse,

l'avis de la commission ?

Lubin. L'expérimentation est fondée sur une logique partenariale de confiance, nous l'avons assez répété. Le fonds d'expérimentation territoriale étant déjà chargé du suivi et de l'évaluation de l'expérimentation, il n'y a pas lieu d'exiger de lui un rapport annuel moral et financier aussi tatillon. Par ailleurs, le fonds bénéficie de moyens limités, y compris en ressources humaines. Il ne s'agit pas d'une grosse entreprise pouvant dédier facilement des ressources à des bilans d'activités fournis.

afin que le fonds soit un acteur de l'expérimentation- essentiellement pour cela, d'ailleurs. Aujourd'hui, l'expérimentation repose sur un pilotage décentralisé et son animation est confiée à un fonds national qui est géré par une association.

La durée de l'expérimentation reste fixée à cinq ans. Il s'agit d'assurer aux territoires, à compter de leur habilitation, la possibilité de bénéficier des modalités de financement tout le temps de leur expérimentation.

il est proposé d'assurer aux territoires, à compter de leur habilitation, la possibilité de bénéficier des modalités de financement tout le temps

L'exhaustivité n'est possible que sur plusieurs années pour mobiliser l'ensemble des demandeurs d'emploi, développer les emplois et les conditions de travail nécessaires, structurer les activités émergentes et non concurrentes. Cinq ans effectifs à partir de l'habilitation

dans l'hypothèse où l'expérimentation devrait ne pas être reconduite, des conventions pourraient demeurer valables, alors même qu'il n'y aurait plus ni fonds, ni habilitation, ni même financement à répartir.

rapidement. Toutefois, si certains territoires devaient entrer plus tard, on saura, au moment où l'on fera le bilan de l'expérimentation, mettre en oeuvre, comme on le fait chaque fois, des dispositions pour permettre à ceux qui sont entrés plus tard

n° 15 rectifié. Ces dispositions introduites en commission des affaires sociales portent atteinte au projet « territoires zéro chômeur de longue durée ». C'est toute la territorialité du projet et la confiance accordée aux territoires pour mener cette expérimentation qui sont mises en danger. En effet, ces nouvelles dispositions visent à imposer une double tutelle : d'une part, une tutelle de Pôle emploi, sur le choix des personnes qui pourront être recrutées dans une EBE, alors même que personne ne le demande- ni les acteurs de terrain ni Pôle emploi -, d'autre part, une tutelle des Direccte, sur le choix des activités développées par les EBE en renvoyant au décret les modalités de ce contrôle. Toute la plus-value territoriale, incarnée par le comité local pour l'emploi, est ainsi niée, alors même que l'ensemble des acteurs saluent cette dynamique territoriale. L'expérimentation repose sur la confiance accordée aux acteurs locaux. C'est la condition de son succès. Cet amendement vise donc à supprimer ces nouvelles tutelles.

au motif qu'elles ne répondent pas exactement aux critères d'éligibilité fixés ? Le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain estime que ce dispositif introduit par la rapporteure de la commission des affaires sociales constitue une sanction disproportionnée et méconnaît la philosophie de l'expérimentation. Il convient donc de le supprimer.

lisez le texte ! À aucun moment, il n'a été fait état d'une tutelle de la Direccte et de Pôle emploi. Je le dis d'autant plus que des mails et des tweets ont circulé, alors que c'est faux. Quand on est rapporteur d'un texte, on est soumis à la pression,

sur les contributions d'assurance chômage et les exonérations de cotisations patronales ; d'autre part, à prévoir l'exonération du bonus-malus des contrats d'insertion conclus avec les structures d'insertion par l'activité économique. à prévoir une application des exonérations de cotisations sans tenir compte de l'effet du bonus-malus, afin de préserver la logique propre à chaque dispositif : effet incitatif du bonus-malus et lisibilité de la réduction du coût du travail résultant des allégements.

exonérations de cotisations patronales. L'objectif de l'article 7 est de garantir l'effet incitatif du bonus-malus, ainsi qu'une meilleure lisibilité de la réduction du coût du travail apportée par les exonérations.

d'emploi. Si nous débattons aujourd'hui du dispositif « territoires zéro chômeur de longue durée », c'est parce qu'il y a un consensus sur le fait que le chômage n'est pas d'abord de la responsabilité des privés d'emploi

des demandeurs d'emploi, le CPF, sera automatique dès lors que la formation sera financée par Pôle emploi ou par la région. Cela signifie que les demandeurs d'emploi seront contraints de puiser dans leurs droits acquis au titre du CPF pour financer une formation dans le cadre de leur retour à l'emploi. Avant la réforme de la formation, un travailleur privé d'emploi pouvait refuser que l'on puise dans son CPF. Cette disposition entretient donc une confusion dangereuse entre ce qui relève de la responsabilité individuelle et ce qui relève de celle de la puissance publique. Elle marque le désengagement de l'État dans l'accompagnement des personnes privées d'emploi, tout en constituant un détournement du CPF, lequel doit rester, selon nous, un outil de formation individuelle pour le salarié. Pour cette raison, nous demandons la suppression de l'article. Quel

désincitatif à l'entrée en formation de la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle. On constate en effet de fortes disparités des conditions d'accès et des niveaux de rémunération, des démarches administratives lourdes et des pertes financières liées à l'entrée en formation. formation. En 2018, pour les 40 % de stagiaires demandeurs d'emploi non indemnisés par Pôle emploi, la rémunération était fixée par un barème qui n'avait pas été revalorisé depuis 2002.

Cet amendement a donc pour objet de mettre en oeuvre la mesure de revalorisation de la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle prévue dans le cadre du plan France Relance.

Madame la ministre, mes chers collègues, il est très bientôt vingt heures et il nous reste douze amendements à examiner.

En effet, l'habilitation définie à l'article 5 permet aux collectivités territoriales, aux EPCI ou aux groupes de collectivités territoriales volontaires de candidater à l'expérimentation pendant trois ans à compter de la date de leur habilitation. Si un territoire est habilité au bout de trois ans, l'expérimentation ne durera effectivement que deux ans. Nous souhaitons prolonger cette durée et la porter à cinq ans.

formation. La législation actuelle, qui limite aux entreprises de moins de cinquante salariés le financement du développement des compétences des salariés, entrave la capacité des SIAE au-delà de ce seuil à mettre en oeuvre de la formation au bénéfice des personnes en parcours d'insertion.

comme en reconversion. Des aménagements pourront être validés d'ici au premier trimestre 2021, en concertation avec les acteurs de l'IAE et de la formation

pour la renforcer que ces dernières sont devenues éligibles à l'accord-cadre national pour la formation des salariés de l'IAE, le PIC IAE, depuis 2020. Des actions de formation à destination des salariés des EBE sont déjà prises en charge,

à Mme Martine Berthet. Cet amendement vise à prolonger de deux ans l'expérimentation du contrat de professionnalisation, afin de permettre aux structures de l'insertion par l'activité économique de s'en saisir.

nous vous proposons de prolonger l'expérimentation relative aux entreprises d'insertion par le travail indépendant (EITI).

vous, madame la rapporteure, le fonds d'indemnisation est mieux à même d'identifier ces particularités. Il nous paraît essentiel de le rappeler, les outre-mer souffrent d'un retard économique persistant en raison, notamment, des difficultés structurelles liées à leur situation géographique et à l'étroitesse de leur marché. Le taux de chômage des territoires ultramarins est parmi les plus élevés de l'Union européenne. Il est au minimum le double de celui de l'Hexagone, voire le quadruple à Mayotte.

nous ne partageons pas toutes les obligations imposées par Mme la rapporteure. Nous regrettons également que certaines exigences ne soient pas- certes, ce n'est pas de votre fait, madame la rapporteure

une véritable chance, d'un point de vue tant économique qu'humain. Les personnes sont sorties de leur isolement social et se sentent reconnues. L'entrée dans l'entreprise à but d'emploi en CDI leur permet de vivre leur quotidien plus sereinement et de se projeter de nouveau dans l'avenir.

proposer des outils complémentaires de pilotage et des expérimentations, tout en gardant comme boussole l'insertion de nos concitoyens les plus éloignés de l'emploi. Le Sénat a fait son oeuvre et ce texte parlementaire est désormais entre les mains de la CMP. La procédure accélérée ayant été engagée, celle-ci

Dans la période d'incertitude que nous connaissons, marquée par des difficultés accrues pour les plus fragiles, son adoption est dans l'intérêt de tous, en particulier des territoires. Ce texte est d'abord un bel objet de lutte en faveur de l'emploi pour tous et de l'égalité des chances. Les deux très beaux outils qu'il renforce appliquent des méthodes complémentaires pour insérer les personnes les plus éloignées de l'emploi. Les SIAE vont voir leurs règles de recrutement

avec les acteurs des structures de l'insertion par l'activité économique et avec l'association Territoires zéro chômeur de longue durée. Pendant sa discussion à l'Assemblée comme au Sénat, un travail constructif a été mené par les députés et les sénateurs de tous les groupes, ce que je tiens à souligner. Les débats ont ainsi permis de mieux répondre aux problématiques des personnes les plus éloignées de l'emploi, en travaillant à leur insertion durable dans l'emploi. Nous avons ainsi oeuvré ensemble, mesdames, messieurs les sénateurs, en faveur d'une relance plus inclusive et de solutions d'accès à l'emploi déployées au coeur des territoires. Je vous en remercie vivement.